dont notre groupe avait demandé l'inscription à l'ordre du jour qui lui est réservé dans le cadre de l'initiative parlementaire. Notre proposition de loi, attendue par des dizaines de milliers d'anciennes agricultrices et d'anciens agriculteurs, avait été adoptée à l'unanimité par la commission des affaires sociales du Sénat.

La Nation leur doit une forme de reconnaissance, de prise en compte de ce grand effort. Le 7 mars dernier, le Gouvernement a agi avec violence en utilisant une procédure rarissime à l'égard d'une initiative parlementaire. Le vote bloqué obligeait le Sénat à se prononcer par un seul vote sur un amendement déposé par le Gouvernement visant à reporter à 2020 la seule éventualité d'une augmentation des retraites agricoles et, dans le même temps, sur le texte dans son ensemble. En clair, soit nous acceptions le renvoi aux calendes grecques de la revalorisation des retraites agricoles, soit nous votions contre notre propre texte ainsi défiguré. Comment ne pas faire le lien entre cet acte autoritaire et les projets de remise en cause des droits des parlementaires dans le projet de loi constitutionnelle à venir ? Monsieur le président, madame la secrétaire madame la ministre des solidarités et de la santé a annoncé officiellement, à l'issue de la séance du 7 mars dernier, qu'elle recourrait de nouveau à la procédure du vote bloqué si le texte était de nouveau présenté au débat sénatorial. À quelques heures de ce débat, pourrions-nous savoir si le Gouvernement entend revenir sur son coup de force, sans le conditionner à tel ou tel compromis que l'on sent de toute façon « piégeux » ? Le Sénat, selon nous, ne peut délibérer ainsi, sous la contrainte.

groupe socialiste et républicain, de la proposition de loi visant à instaurer un régime transitoire d'indemnisation pour les interdictions d'habitation résultant d'un risque de recul du trait de côte, présentée par Mmes Françoise Cartron et Laurence Harribey et par M. Philippe Madrelle

déposée il y a quelques semaines, cette proposition de loi dont nous avons à débattre aujourd'hui vise à prévoir un régime d'indemnisation pour les interdictions d'habitation résultant d'un recul du trait de côte.

Cette affaire, que nous connaissons désormais trop bien dans les assemblées parlementaires, est inédite, exceptionnelle et injuste. Elle est aussi devenue inextricable, car, hélas, à ce jour, aucune solution n'a pu être trouvée.

et ce- faut-il le rappeler ? -, sans aucun dédommagement. Le problème est désormais connu bien au-delà du sud du Médoc. Tout le monde a en tête l'image de cet immeuble à l'abandon, face à la mer.

ubuesque perdure, car l'interdiction effective d'habiter le bâtiment ne vaut pas expropriation, ce qui aurait donné lieu à une indemnisation à hauteur du prix de En effet, conformément au code de l'environnement, l'expropriation donne lieu à une indemnisation si, et seulement si, il existe une menace grave pour la vie humaine, ce qui n'est pas le cas des risques d'érosion côtière. En conséquence, en l'absence d'expropriation, le fonds dit « Barnier », qui permettrait d'indemniser les copropriétaires, n'a pu être mobilisé.

Après quatre années de contentieux avec l'État, dont je rappelle que la responsabilité est totalement engagée, il est urgent de répondre légalement à cette problématique, qui devient pour les personnes concernées proprement insoutenable. Depuis quatre ans, onze des copropriétaires sont décédés.

Pourquoi cette situation perdure-t-elle ? Disons-le très clairement : si cet enfer est encore aujourd'hui devant nous, c'est par manque d'efficacité, par manque de volonté et du fait de tergiversations politiques.

la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable l'a parfaitement rappelé en commission le 16 avril dernier : « Ce texte reprend à l'identique un article de la proposition de loi de notre collègue Michel Vaspart que le Sénat a adoptée en janvier dernier

je vous demande, madame la secrétaire d'État, d'utiliser ce véhicule législatif pour la déposer par voie d'amendement et la faire entériner par votre majorité à l'Assemblée nationale. Nous ne demandons que cela, et tout le monde retiendra qu'il s'agit d'une réponse collective. Il eût d'ailleurs été intéressant que tous les groupes politiques qui se sont penchés sur cette question soient associés à la réflexion, afin d'envisager une sortie de crise. La concertation n'a pas été au rendez-vous, mais une sortie par le haut est toujours possible. En effet, il ne faudrait pas que s'installe l'impression que des solutions sont trouvées facilement pour les plus riches dans d'autres lieux et dans d'autres textes, alors que, pour certains, il faut toujours attendre. C'est pourquoi nous faisons de cette situation un symbole non seulement environnemental, mais aussi, et avant tout, social et humain. Car cela commence à faire beaucoup- beaucoup de textes, beaucoup d'unanimités -pour bien peu d'avancées. Les propriétaires en ont assez du manque d'informations, assez d'entendre parler de rapidité et d'équité, assez de savoir que, chaque jour qui passe, leur responsabilité est engagée en cas d'accident consécutif à la chute de l'immeuble, de l'immeuble, assez d'être assimilés à des privilégiés alors qu'ils sont le plus souvent des retraités modestes épuisés moralement et physiquement, qu'ils ont pour beaucoup investi toutes leurs économies et qu'ils se sont parfois engagés jusqu'en 2030 pour le remboursement de leur prêt.

Début 2014, nous avons été expulsés de cet appartement par un arrêté de péril. [ ...] Depuis, c'est un calvaire, un cauchemar que nous vivons. Outre l'enfer d'avoir été expulsés de chez nous sans aucune aide proposée, sans aucun accompagnement. [ ...] « Aujourd'hui, je travaille, mais je dois faire face aux frais d'un logement de 656 euros de loyer hors charges, je dois rembourser un crédit de 550 euros pour l'appartement de Soulac-sur-Mer hors charges que je ne peux pas habiter, le tout avec un salaire de 1 800 euros. Si je rajoute les frais d'énergie, les impôts, les frais pour aller travailler, il me reste entre 100 et 200 euros pour vivre et faire vivre ma famille. [ ...] « Drôle de traitement pour des citoyens pourtant exemplaires, majoritairement des gens simples. Nous avons été obligés de faire une action en justice dans ce dossier, bien à contrecoeur, rien ne se passant. Nous sommes à bout nerveusement, physiquement, intellectuellement. À tout cela s'ajoute l'humiliation subie par le fait que dans la même ville de Soulac-sur-Mer, à deux kilomètres de chez nous, a été protégée à grands frais une zone pavillonnaire.

La proposition de loi que nous examinons aujourd'hui porte sur un sujet bien connu de certains d'entre vous, puisque son article unique figurait déjà dans la proposition de loi portant adaptation des territoires littoraux au changement climatique, qui n'avait pas pu aboutir lors de la précédente législature, compte tenu de la suspension des travaux parlementaires. Ces mêmes dispositions ont ensuite été reprises dans la proposition de loi relative au développement durable des territoires littoraux, déposée en septembre 2017 au Sénat par notre collègue Michel Vaspart et adoptée par notre assemblée en janvier dernier. Vous le voyez, madame la secrétaire d'État, le Parlement est constant sur ce sujet, et il est plus que temps que le Gouvernement reconnaisse enfin l'urgence qu'il y a à le traiter.

-, dans lequel la responsabilité de l'État est évidente et son inaction préjudiciable aux copropriétaires de l'immeuble du Signal. Dans le cadre de l'ancienne mission interministérielle pour l'aménagement de la côte Aquitaine, active des années 1960 à la fin des années 1980, un grand programme de constructions était prévu à Soulac-sur-Mer en Gironde, sur 19 hectares de terrain. Environ 1 200 logements devaient être construits le long du front de mer, ainsi qu'un boulevard de deux fois trois voies, un établissement de thalassothérapie et un hôtel de luxe. Ce projet n'a jamais vu le jour, l'aménageur retenu par les pouvoirs publics ayant déposé le bilan. Seul un immeuble de 78 logements, le Signal, a été construit, pour le malheur aujourd'hui de ses propriétaires. En 1967, il se situait à plus de 200 mètres du rivage. Les habitants présents depuis l'origine rapportent même que l'on peinait à voir l'océan Aujourd'hui, Le Signalest à moins de 10 mètres du rivage et menace de tomber. Les propriétaires, expulsés en trois jours, mais non expropriés, depuis 2014, par arrêté du maire de Soulac-sur-Mer, demandent tout simplement à être indemnisés pour leur bien. bien. La situation des propriétaires du Signal est ubuesque, parce que c'est l'État qui a décidé de lancer une opération d'aménagement à Soulac-sur-Mer. C'est l'État qui a accordé le permis de construire, et c'est l'État qui, à cette époque, ne pouvait ignorer que plusieurs immeubles du front de mer étaient déjà tombés de la falaise dunaire dans les années 1930. La situation actuelle relève donc de la responsabilité de l'État. Ce dossier est également kafkaïen, parce que la situation juridique des propriétaires est absurde. Ils ont engagé une procédure contentieuse dès 2013, d'abord pour demander au maire et aux représentants de l'État dans le département de mettre en place un enrochement autour de l'immeuble. Cela leur a été refusé au motif que le coût de protection s'élevait à 17 millions d'euros, ce qui dépassait largement la valeur de l'immeuble, estimée à 10 millions d'euros, le tout sans prendre en compte le risque du recul du trait de côte. L'action contentieuse des propriétaires Barnier. En 2014, le ministre de l'écologie, Philippe Martin, s'était rendu sur place avec le préfet et avait promis « un règlement rapide et équitable ». Les deux objectifs de rapidité et d'équité ne sont toujours pas atteints quatre ans plus tard. À l'heure actuelle, la situation est inextricable. En effet, un arrêté portant ordre d'évacuation et interdiction d'occupation de l'immeuble a été publié le 24 janvier 2014 par le maire de Soulac-sur-Mer, au titre de ses compétences de police administrative. Les habitants sont donc privés de la jouissance de leur bien et des fruits de leur propriété, tout en restant propriétaires ; ils pourront par ailleurs voir leur responsabilité engagée en cas d'accident consécutif à la chute de l'immeuble. L'affaire du règlement de cette procédure est pendante devant le Conseil d'État et devrait intervenir au mois de juin prochain, le Conseil constitutionnel ayant rendu sa décision sur la question prioritaire de constitutionnalité, soulevée par les propriétaires, relative aux dispositions de l'article L. 561-1 du code de l'environnement le 6 avril dernier, en écartant les griefs tirés de la méconnaissance du principe d'égalité devant la loi et du droit de propriété. Une fois la décision du Conseil d'État rendue, les propriétaires pourront ultimement saisir la Cour européenne des droits de l'homme. À ce stade, l'administration refuse toujours d'accéder à la requête des propriétaires visant à obtenir une indemnisation le fonds Barnier, pour deux motifs d'abord, parce que l'érosion dunaire n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 561-1 du code de l'environnement, qui définit le champ d'intervention du fonds Barnier

Ensuite, au-delà du contenu de ce dossier, la dimension humaine du sujet est essentielle et me paraît très insuffisamment mentionnée dans le débat public. On a entendu bien des choses sur les propriétaires du Signal, qui seraient des nantis, des privilégiés, et qui devraient assumer sans se plaindre les conséquences de leur désir de vivre au bord de l'eau. Je souhaite couper court à ces représentations, car la majorité d'entre eux sont en réalité des personnes séduites par le projet initial, mais de condition modeste, et aujourd'hui très éprouvées moralement et physiquement par la longueur des procédures et un manque d'informations sur la réalité des initiatives conduites pour leur apporter une solution. Certains ont investi toutes leurs économies et doivent en plus, cela a été rappelé, continuer à rembourser leur dette jusqu'en 2020, 2025, voire 2030 ; d'autres d'autres ont dû se reloger et acquittent un loyer ; tous continuent d'assumer les frais de syndic de copropriété, les assurances et le coût d'une procédure longue et coûteuse pour se défendre. Les frais d'avocats s'élèvent à 100 000 euros depuis 2012, d'après leurs représentants. ailleurs, depuis quatre ans, date de l'évacuation, onze propriétaires sont décédés. La question des successions est alors apparue comme un nouveau problème pour leurs descendants, qui sont en contact avec l'administration fiscale pour estimer la valeur de la transmission, ajoutant du découragement Quant à l'immeuble, il a été vandalisé et occupé de façon irrégulière en dépit de nombreuses plaintes des propriétaires. Il est en très piteux état, sa protection par la commune n'est pas suffisamment assurée à ce jour, alors même que cette dernière pourrait voir sa responsabilité engagée en cas d'accident.

Si le recul du trait de côte s'impose comme un phénomène commun à de nombreux territoires et s'il nécessite une approche intégrée et globale, sans doute davantage dans une logique d'acquisition que d'indemnisation, le cas du Signal est inédit est injuste. Cette situation a trop duré, je le dis fermement. Selon l'Observatoire de la côte Aquitaine, le trait de côte recule de 2,5 mètres en Gironde chaque année et de 1,7 mètre dans les Landes. Dans le cas du Signal, le recul du trait de côte est de 5 à 7 mètres par an en moyenne, recul accentué notamment par la présence d'une digue à proximité, qui protège le le quartier de l'Amélie à Soulac-sur-Mer et qui a tendance, de plus, à accélérer les courants et à empêcher le sable de se stabiliser. Si nous sommes d'accord sur la nécessité de régler le problème de l'indemnisation et de la propriété de l'immeuble,

à rendre éligibles les propriétaires de l'immeuble du Signal à une indemnisation rétroactive par le fonds de prévention des risques naturels majeurs, dit « fonds Barnier », créé en 1995. Nous Nous devons également éviter qu'une telle situation ne se reproduise. C'est pourquoi il est fondamental d'inscrire rapidement dans les textes une obligation d'information préalable à l'acquisition d'un bien proche proche du rivage, pour que les futurs propriétaires de ce type de biens aient pleinement conscience du risque de recul du trait de côte. Madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, sur le fait qu'un amendement du Gouvernement serait nécessaire pour établir clairement un transfert de propriété. En l'état, le dispositif permettra uniquement d'indemniser les propriétaires. Il faut conclure, ma chère collègue. Les charges de démolition et de désamiantage leur incomberont également.

J'espère sincèrement que nous pourrons trouver collectivement une réponse rapide. C'est indispensable. Sous le bénéfice de ses observations, la commission vous invite, mes chers collègues, à adopter le présent texte sans modification. La parole

Monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs,

plus que jamais impératif de repenser l'élaboration de nos politiques publiques et d'anticiper les effets du changement climatique, pour imaginer et travailler ensemble au littoral de demain.

loi pose de nouveau et à juste titre la question des modalités d'indemnisation des propriétaires de biens menacés par ces phénomènes d'érosion côtière. Le trait de côte est mobile

en tenant compte des conséquences du changement climatique. Au contraire des crues ou des séismes, qui surviennent de façon aléatoire et renouvelée, le recul du trait de côte, même s'il est inéluctable, ne peut être

Gironde. Confirmant la position de l'État sur les conditions d'éligibilité à l'expropriation pour les risques naturels majeurs, le Conseil constitutionnel considère que l'érosion côtière ne permet pas de déclencher une expropriation au titre d'un risque naturel majeur. Cette spécificité du phénomène d'érosion appelle donc de nouvelles solutions d'ensemble et structurantes. Elle suppose, en premier lieu, l'adaptation de nos territoires littoraux menacés. Comme je le détaillais déjà en janvier dernier, deux mesures me semblent aller en ce sens. D'abord, je suis convaincue qu'il est nécessaire d'offrir aux collectivités compétentes des outils adaptés en matière d'aménagement du territoire. Ensuite, il est également nécessaire de faire évoluer le cadre juridique existant pour mieux prendre en compte la temporalité de ce phénomène dans les documents d'urbanisme.

madame la sénatrice, mais nous voulons un texte global parce que lui seul permettra de traiter à la fois de la question de l'anticipation des phénomènes d'érosion côtière, par le biais, notamment, d'une description et d'une intégration dans les documents d'urbanisme par les acteurs compétents, de la question de l'indemnisation des biens existants qui ont été ou seront atteints à court terme par l'érosion et, enfin, de la question de relocalisation, de la conception et du déploiement de projets dans les territoires préservés à plus long terme.

je partage avec vous le souci et l'exigence de trouver au plus vite une réponse équilibrée afin de mettre un terme à cette situation, qui est, il est vrai, comme vous l'avez souligné, très difficile pour certains des copropriétaires. Le ministre d'État a également eu l'occasion d'exprimer sa préoccupation sur cette question et sa volonté d'identifier rapidement des solutions pratiques pour cette situation spécifique et particulière.

Nous avons d'ores et déjà demandé au préfet de région d'organiser des opérations de désamiantage de l'immeuble pour prévenir, sans attendre, les risques pour la santé publique et l'environnement. Vous pouvez aisément l'imaginer, si l'immeuble venait à s'effondrer, l'amiante contaminerait tout l'environnement. Il est en effet impératif d'agir vite sur cette question, et je sais par ailleurs que vous partagez ici la nécessité d'avoir une approche globale en faveur d'une gestion intégrée du trait de D'aucuns pensent peut-être qu'elle pourra intervenir dans un second temps, après avoir réglé la situation des copropriétaires du Signal. Pour ma part, je considère que la question de l'indemnisation ne peut pas être traitée indépendamment. Elle doit faire partie d'un tout : il faut régler la question de l'acquisition de l'immeuble pour pouvoir le détruire et apporter aux autres territoires l'ensemble des outils nécessaires à la transformation de nos littoraux. Cela suppose que les collectivités intéressées soient parties prenantes des décisions prises à court et long termes. C'est pourquoi le Gouvernement émet un avis défavorable sur la proposition de loi qui nous est aujourd'hui

Celui-ci devrait nous permettre d'atteindre dans les meilleurs délais l'objectif ciblé et légitime que nous défendons tous, à l'instar de Mmes les sénatrices Cartron et Tocqueville.

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, madame la rapporteur, mes chers collègues, en début d'année, nous avions discuté en ce lieu d'une proposition de loi tendant en partie à réviser la loi Littoral, dans une perspective globale d'aménagement des territoires littoraux. Beaucoup d'entre nous dans l'hémicycle avaient peur d'ouvrir la boîte de Pandore : les avantages d'un tel assouplissement auraient pu avoir des effets pervers. Nous étions tous d'accord pour reconnaître le bienfait de la loi Littoral, mais nous ne placions pas le curseur au même endroit. Il est nécessaire de lever les blocages, mais pas à n'importe quel prix ni dans n'importe quel cadre. Néanmoins, si l'article 9 nous opposait, l'article 3 faisait plutôt consensus : il s'agissait de résoudre la situation des propriétaires de l'immeuble Le Signal à Soulac-sur-Mer. La question du recul du trait de côte ne fera peut-être pas la une des journaux, pourtant cette problématique, au-delà de Soulac-sur-Mer, concerne aujourd'hui beaucoup de monde, et elle en concernera encore beaucoup plus demain. Rappelons qu'un Français sur dix vit sur le littoral et que les départements d'outre-mer comptent près de cent dix communes littorales. Pour bien comprendre les enjeux de la question du recul du trait de côte, il faut avoir en tête deux choses que l'on ne connaissait pas il y a trente ans au moment de la loi Littoral. Premièrement, l'érosion connaît des phases d'accélération dues au réchauffement climatique dont nous sommes responsables. Deuxièmement, l'érosion est moins prévisible qu'on ne le pensait : sa survenue s'apparente parfois à une catastrophe naturelle. Vous le savez, mes chers collègues, nous ne pouvons pas faire des lois pour régler chaque cas particulier. Mais nous ne pouvons pas non plus, au motif de chercher des dispositifs élaborés et globaux mais qui mettent plusieurs années à être opérationnels, refuser de regarder en face les situations dramatiques que vivent nos concitoyens. L'équilibre entre la hauteur de vues et la réalité concrète, avec ses souffrances réelles, est parfois précaire. Aussi, mes chers collègues, mon groupe soutient avant tout une réflexion globale et collective sur les enjeux liés au littoral. Nous devons en priorité développer une culture de la prévention qui anticipe les risques liés au dérèglement climatique. Mais, considérant que la problématique du trait de côte se présente sous un jour que ne pouvait pas encore connaître le législateur au moment du vote de la loi Littoral, considérant que la dimension de catastrophe naturelle liée à l'accélération de l'érosion justifie la mobilisation du fonds Barnier et, enfin, considérant que la situation de l'immeuble Le Signal n'a que trop durer,

en place un régime transitoire d'indemnisation pour les interdictions d'habitation résultant d'un risque de recul du trait de côte. Il s'agit de la troisième tentative avec, notamment, l'adoption en première lecture par notre assemblée, le 30 janvier dernier, de la proposition de loi relative au développement durable des territoires littoraux, qui restera sans suite. Il y a urgence, madame la secrétaire d'État, et c'est la responsabilité de l'État de trouver une solution concrète à cette situation. Réglons d'abord ce problème et- chiche !-comme vous l'avez dit, travaillons sur un texte plus vaste. Il est essentiel de gommer aujourd'hui cet angle mort du dispositif de prévention des risques naturels majeurs. Rappelons que l'État a autorisé et supervisé la construction d'un immeuble sur une zone où le risque n'était pas inenvisageable. Pire, le droit censé protéger les citoyens est ici lacunaire, l'érosion dunaire n'étant pas prise en compte au titre des risques naturels indemnisés par le fonds Barnier. Ainsi délogés sans indemnisation et après plusieurs années de procédures judiciaires au cours desquelles ils ont épuisé tous les recours, ces hommes et ces femmes se sentent abandonnés par les pouvoirs publics. Il est de notre rôle de législateur de régler ce problème et de débloquer une indemnisation légitime et de bon sens. Nous sommes ainsi favorables à cette proposition Par ailleurs, ce cas d'espèce nous rappelle l'importance de la loi Littoral quant à l'aménagement de nos côtes. Nous ne pouvons plus nier le recul du trait de côte et déléguer la gestion de son impact aux générations futures. Une réflexion aurait été nécessaire sur les possibilités d'urbanisation dans des zones aussi proches du littoral et leur relocalisation sans pour autant défigurer les terres par une urbanisation discontinue et consommatrice de terrains agricoles ou naturels. Cela doit également nous interpeller sur l'ensemble des situations similaires présentes tout le long de notre façade maritime. Il nous faut envisager un mécanisme d'indemnisation plus large, par équité envers les autres citoyens lésés par le recul du trait de côte. Progressivement, les missions du fonds Barnier sont élargies, mais les moyens de ce dernier sont réduits chaque année. La loi de finances pour 2018 a également prévu le plafonnement de la taxe dévolue au fonds Barnier à hauteur de 137 millions d'euros, réaffectant ainsi près de 90 millions au budget général. Ce montant est très inférieur aux dépenses constatées ces dernières années, équivalant à 178 millions d'euros. De manière plus générale, le budget consacré aux risques hydrauliques et naturels est en constante régression. À ce titre, la discussion de la proposition de loi relative au développement durable des territoires littoraux avait donné lieu à une discussion intéressante qu'il faudra reprendre rapidement, car la situation est urgente : en cinquante ans, le territoire français a rétréci de 2 600 hectares, l'équivalent de 3 600 terrains de football, témoin concret de l'ampleur et de la gravité du réchauffement climatique, qui est bien un défi d'aujourd'hui et non de demain. Au-delà de ces aspects plus généraux, nous proposons de voter en faveur de ce texte et espérons vivement que ce travail parlementaire puisse aller à son terme. Bravo

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, monsieur le président de la commission, madame la rapporteur, mes chers collègues, c'est aujourd'hui la troisième fois que nous examinons dans cette assemblée un texte permettant de réparer l'injustice que connaissent les habitants de l'immeuble Le Signal à Soulac-sur-Mer. Je tiens à remercier ma collègue Françoise Cartron, à l'origine de cette proposition de loi, et la rapporteur Nelly Tocqueville pour leur persévérance en faveur de la résolution de cette situation qui n'a que trop duré. Ce texte entend en effet répondre à une urgence, alors même que la situation de l'immeuble Le Signal et de ses copropriétaires nous est désormais familière. Lors de sa construction, en 1967, cet immeuble était éloigné de l'océan de plus de 200 mètres. Aujourd'hui, de tempête en tempête, le trait de côte n'est plus qu'à quelques mètres. Depuis 2014, les habitants ne peuvent plus occuper les lieux, mais aucun dispositif d'expropriation permettant leur indemnisation n'a pu être mis en oeuvre. Nous regrettons tous cet état de fait et les difficultés dans lesquelles se trouvent les copropriétaires. Le Sénat a déjà voté deux propositions de loi intégrant une disposition en réponse à cette situation. Cela a permis de mettre en évidence un consensus sur la mise en place d'un régime transitoire d'indemnisation pour les interdictions d'habitation résultant d'un risque du recul du trait de côte. De plus, la commission des lois avait apporté des modifications au texte initial afin d'éviter que l'équilibre financier du fonds Barnier ne soit remis en cause, et je le salue de nouveau. Or, malgré ce consensus et l'importance des enjeux, la proposition de loi relative au développement durable des territoires littoraux reste inexplicablement bloquée par la majorité de l'Assemblée nationale. La mer monte, la plage disparaît, mais le texte, lui, pendant ce temps, s'ensable. C'est donc pour cesser de perdre un temps précieux que l'article 3 de cette proposition de loi, initiée par notre collègue Michel Vaspart, est ici intégralement la mobilité et l'aménagement, montrent que de plus en plus d'habitations seront touchées par ce phénomène, et l'indemnisation des propriétaires sera au coeur du problème. N'en déplaise aux sceptiques, le changement climatique est une réalité d'ores et déjà visible. La montée du niveau des océans ainsi que l'aggravation de la fréquence et de l'intensité des tempêtes qui en résultent auront un impact important sur nos côtes. Il est donc temps de se saisir de ces problèmes et d'y apporter au plus tôt une réponse appropriée. Mes chers collègues, le groupe UC votera cette proposition de loi, car celle-ci répond à un problème urgent, tout en étant symptomatique des effets de politiques d'aménagement du littoral que nous ne pouvons plus tolérer. Souhaitons que nos collègues du Palais-Bourbon, enfin sensibles à la détresse matérielle et humaine des habitants de l'immeuble Le Signal comme à la prégnance des enjeux auxquels font face les espaces littoraux, adoptent au plus vite cette proposition de loi, mais aussi celle dont elle est issue. Nos concitoyens, nos paysages et notre économie le méritent. Alain Cazabonne, sénateur du groupe Union Centriste, compte d'ailleurs évidemment sur une large adoption de ce texte.

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, monsieur le président de la commission, madame la rapporteur, mes chers collègues, je ne surprendrai probablement personne en disant que le groupe Les Indépendants- République et Territoires votera évidemment ce texte, car il vient en soutien de la proposition de notre de notre collègue et des explications de Mme la rapporteur qui a très bien rappelé la situation. La plupart des groupes qui se sont prononcés depuis le début de la discussion générale vont dans ce sens ; nous sommes donc tout à fait solidaires de cette position. Je suis moi-même issu d'un département littoral qui souffre de l'érosion, dans des conditions

notre littoral dans la partie que l'on appelle « le hâble de Ault » : la mer attaque les falaises de Ault et plusieurs rues de Ault-Onival, qui est une station balnéaire, ont dû être interdites à l'habitation. Ce sont donc des sujets que nous connaissons bien.

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, madame la rapporteur, mes chers collègues, en deux ans, c'est la troisième proposition de loi que nous examinons ayant pour objet d'utiliser le fonds Barnier afin de résoudre le problème de l'immeuble Le Signal. Alors que des textes plus généraux sont encore dans les tuyaux de la machinerie législative, mais risquent fort de ne pas aboutir pour cause d'ouverture de la boîte de Pandore de la loi Littoral, le texte présenté ce jour a le mérite de se limiter au Signal : cette fois-ci, c'est clair.

Répondant à l'urgence aujourd'hui médiatisée de la perte des économies de ces propriétaires d'appartements avec vue imprenable sur la mer, ce texte prévoit de créer un usage dérogatoire du fonds Barnier pour que les copropriétaires concernés puissent bénéficier d'une indemnisation de leurs biens à hauteur de 75 % de leur valeur.

tout simplement reconnaître la responsabilité de l'État dans la délivrance du permis de construire. Plutôt que d'avoir un débat très général, on devrait peut-être simplement se dire que l'État n'aurait pas dû délivrer ces permis de construire ;

Considérant que cette proposition de loi offre les garanties nécessaires à une application très circonscrite du fonds Barnier au cas de l'immeuble Le Signal, une majorité du groupe du RDSE votera ce texte, alors que l'autre partie du groupe- c'est aussi légitime -considérant qu'il pose trop de problèmes juridiques,

le sujet qui nous réunit cet après-midi appelle- enfin ! -une réponse du Gouvernement, alors qu'il est sollicité pour la troisième fois sur l'éligibilité de l'indemnisation du recul du trait de côte au titre du fonds Barnier. Mes collègues Françoise Cartron, auteur de la présente proposition de loi, et Nelly Tocqueville, rapporteur, ont parfaitement restitué le contexte avant moi : il s'agit de traiter le cas particulier des propriétaires de l'immeuble Le Signal construit à Soulac-sur-Mer, en Gironde, dans les années impactés par une interdiction définitive d'habiter ou d'occuper les lieux prise en raison de l'érosion du trait de côte, tant et si bien que l'immeuble est devenu inhabitable depuis de nombreuses années déjà, sans qu'ils aient été expropriés ni indemnisés,

et la proposition de loi relative au développement durable des territoires littoraux, que j'ai déposée avec mes collègues Retailleau et Bas et qui fut largement adoptée par le Sénat en séance publique en janvier dernier.

Les mois passent, et les propriétaires, pour la plupart de modestes retraités, attendent désormais seulement, si j'ose dire, une indemnisation. Face à cette situation, vous nous avez opposé un refus en janvier, en nous disant que l'érosion dunaire n'entrait pas dans le champ d'application de l'article L. 561-1 du code de l'environnement. Il est par ailleurs pris acte du sort de la question prioritaire de constitutionnalité déposée par le Conseil d'État,

... Certes, la création de ce groupe de travail sera peut-être un progrès puisque le recul du trait de côte est général : il appelle une réflexion globale et des solutions de principe et pérennes de façon à anticiper ces difficultés pour les propriétaires, les élus et les professionnels de la mer. Mais s'agissant du cas particulier de l'immeuble Le Signal, vous comprendrez, madame la secrétaire d'État, qu'il ne soit pas possible d'attendre. C'est d'ailleurs à l'unanimité que la commission a adopté ce texte le 18 avril dernier, afin de prévoir ce cas éligible au fonds Barnier. J'y suis personnellement plus que favorable et je soutiens fortement cette proposition de loi discutée dans la niche réservée au groupe socialiste et républicain. Il est des sujets, madame la secrétaire d'État, qui transcendent et qui devraient transcender les clivages politiques, et c'en est

C'est un message que je m'efforce de faire passer depuis mon élection au Sénat en 2014. Les élus locaux du littoral comme les associations de propriétaires dans ce domaine ne font pas de politique, ils sont pragmatiques il n'est pas question de porter atteinte à l'environnement, il est seulement question, si j'ose dire, de trouver des solutions pragmatiques utiles à nos concitoyens et aux élus qui les représentent, sans dogmatisme. que le ministre, les secrétaires d'État et les hauts fonctionnaires du ministère soient dans le même état d'esprit. Vendredi dernier encore, je me suis rendu à Plestin-les-Grèves, dans mon département des Côtes-d'Armor, sollicité par une famille sommée de détruire sa maison, détient pourtant un permis de construire en bonne et due forme, une maison écologique à énergie positive construite dans une dent creuse. J'ajoute que la mairie s'est vu refuser l'extension de sa zone d'activité, alors qu'elle est en continuité de celle qui existe déjà. Nous allons là au-delà de la loi de 1986. Excès de zèle ou parapluie inutile ? Madame la secrétaire d'État, cela n'est plus supportable et les élus locaux ne le supportent plus. Aujourd'hui, si le Gouvernement continue de faire la sourde oreille, ce sera non pas une erreur, mais une faute impardonnable. Sur tous ces points, la position du Gouvernement doit être clarifiée, pour que chacun soit au clair et prenne ses responsabilités. Comment comprendre la remise à plus tard et la création de groupes de travail, alors que le travail a été fait par les représentants du peuple, notamment par le Sénat ? Pour en revenir au Signal, je voterai cette proposition de loi sans aucune réserve, et c'est aussi la position de mes collègues du groupe Les Les propriétaires du Signal ne peuvent plus attendre. J'aimerais vous convaincre aussi de l'urgence à ouvrir clairement le sujet de la clarification de la jurisprudence sur la loi Littoral, en lien avec notre droit de l'urbanisme.

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, madame la rapporteur, mes chers collègues, mon intervention

Les planificateurs ne sont pas allés au bout de l'aménagement, car, comme par hasard, ils n'avaient pas prévu le recul du trait de côte. Le droit est rarement en amont des faits. Depuis quatre ans, les propriétaires se voient interdire l'accès à leur bien, sans pour autant avoir été expropriés en droit, au motif que l'article L. 561-1 du code de l'environnement n'établit pas de lien formel entre l'érosion côtière et la menace grave pour la vie humaine. Par voie de conséquence, impossible pour eux d'être indemnisés par le fonds Barnier.

Or un vide juridique est fait pour être comblé. Tel est l'objectif de cette proposition de loi, d'une clarté à toute épreuve et d'une grande simplicité.

sortiront grandies ! La discussion générale est close. Nous passons à la discussion du texte de la commission.

loi qui s'inscrit pleinement dans l'esprit de la loi Barnier ? J'ai bien compris que, en s'appuyant sur le code de l'environnement, le Gouvernement considère

madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, cette proposition de loi, qui certes a un caractère exceptionnel, permet d'envoyer un message fort sur le registre du symbolique. L'évolution du trait de côte est une préoccupation constante des riverains, qui se perçoivent comme des victimes potentielles. Je puis vous assurer que les porter à connaissance des zones rouges définies dans les plans de prévention des risques de submersion marine par les DREAL

pour faire face aux indemnisations. Certes, il faut une approche globale ; mais le mieux est souvent l'ennemi du bien. Cette proposition de loi, bien que de portée limitée, constitue une avancée.

! J'entends que, d'un point de vue technique, technocratique, il est très compliqué de trouver une solution en s'appuyant sur tel texte, amendement, contre-texte ou autre. Mais le résultat,

de devoir à nouveau discuter de cette question, que le Sénat a déjà tranchée à plusieurs reprises ! Pourquoi sommes-nous dans cette situation ? Tout

et celui qui l'a précédé n'ont pas voulu prendre leurs responsabilités pour traiter ce problème. Il y a, bien sûr, le problème de l'immeuble Le Signal, symptomatique des difficultés que nous rencontrons du fait du recul du trait de côte ; mais il n'épuise pas le sujet.

de la construction dans les dents creuses, sans oublier l'évolution du fonds Barnier et de ses financements. Il n'est pas admissible que, chaque année, le gouvernement détourne pour le budget de l'État une partie du produit de ce fonds, ... Voilà ! ... qui vient tout de même des assurances Alors que nous avons les moyens d'agir avec le fonds Barnier, on le dégonfle artificiellement pour utiliser cet argent à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été institué ! Je préférerais de beaucoup qu'on élargisse les possibilités de financement du fonds Barnier et que l'on traite l'ensemble des questions, y compris celles qui sont relatives à la construction,

les textes que nous avons votés ! Je lui dis : n'ayez pas d'amour-propre d'auteur, car le problème est de régler les difficultés qui assaillent de très nombreux Français devant le recul du trait de côte

la responsabilité de l'État est engagée, il faut une réponse rapide. Il ne faut surtout pas mélanger la situation du Signal et les réponses à l'évolution du trait de côte liée au réchauffement climatique. Évidemment ! Si vous faites les deux à la fois, vous n'arriverez à rien

cours de droit constitutionnel, mais ce n'est pas parce qu'on n'est pas d'accord avec un texte voté par le Sénat qu'on ne doit pas l'inscrire à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale ... Les députés peuvent modifier un texte qui ne correspond pas aux souhaits de la majorité de l'Assemblée nationale et du Gouvernement.

nous poursuivrons ensemble le travail. Nous continuerons à travailler pour que les copropriétaires du Signal finissent par avoir gain de cause. Nous le leur devons ! C'est une simple question d'honnêteté, mais aussi une question d'assistance à personne en danger ! L'ordre

le 2 avril 2013, celui-là même qui était parfois assis, dans cet hémicycle, au banc du Gouvernement, chargé quelques mois plus tôt par le Premier ministre de redresser les comptes publics et de lutter contre l'évasion fiscale, celui-là même qui, devant la représentation nationale, avait menti en niant catégoriquement avoir jamais détenu de compte bancaire à l'étranger, ce jour-là, le 2 avril 2013, Jérôme Cahuzac reconnaissait détenir des fonds non déclarés sur un compte bancaire, en Suisse, puis à Singapour. Nous le savons, l'histoire de la lutte contre la fraude et la corruption progresse souvent par crises. Crises de confiance, d'abord. Ce coup porté à la démocratie, ébranlant l'opinion, a agi comme un électrochoc et ouvert la voie à des avancées majeures dans cette lutte et dans la transparence de la vie publique.

grâce à l'instauration de ces nouvelles institutions, désormais incontournables. Mais nous devons aujourd'hui aller plus loin. Nous l'avons vu lors de la campagne présidentielle de 2017, elle aussi marquée par une profonde crise. Les scandales qui l'ont rythmée sont à l'origine des lois sur la transparence de la vie politique de septembre 2017. Ils nous rappellent à tous qu'on ne parvient jamais au

des procédures fiscales, en vertu duquel l'auteur d'une infraction fiscale ne peut être poursuivi que sur plainte de l'administration et, au surplus, sous réserve d'un avis conforme de la commission des infractions fiscales, la CIF. Nous le connaissons dans cet hémicycle,

le cas en mars 2016, avec l'adoption d'un amendement déposé par notre collègue Éric Bocquet, ou encore plus récemment, en 2017, avec l'adoption d'un amendement proposé par notre collègue Éliane Assassi. Par deux fois, l'Assemblée nationale s'est engagée dans la même démarche. Pourtant, en 2017, décision a été prise de se donner un temps de réflexion supplémentaire. Nos collègues députés ont créé une mission d'information commune sur les procédures de poursuite des infractions fiscales, commission qui rendra son rapport dans les jours à venir.

Cette anomalie est largement dénoncée, au-delà des travées du Sénat. Ainsi Éliane Houlette, procureur de la République financier, devant l'Assemblée nationale voilà quelques jours, a dénoncé la situation en ces termes le verrou bloque toute la chaîne pénale. Il empêche la variété des poursuites et constitue un obstacle théorique, juridique, constitutionnel et républicain, en plus d'être un handicap sur le plan pratique.

De nombreuses ONG- j'ai cité Transparency International, mais on peut ajouter Oxfam, Sherpa ou Anticor -rappellent depuis plusieurs années la désuétude de ce dispositif. Il est donc plus que temps d'y mettre fin, car il est indispensable que la justice puisse se saisir en toute transparence des infractions fiscales, en particulier des plus graves. Nous regrettons que le Gouvernement ait fait le choix de l'immobilisme, en n'intégrant pas cette disposition dans le projet de loi présenté le 28 mars dernier et dont nous aurons à débattre dans quelques semaines. Effectivement,

instants. Il invoque des motifs d'efficacité et de compétence fiscale d'une haute technicité. Ce point de vue, pourtant, ne tient compte ni du gain d'efficacité indéniable rendu possible par la Cour de cassation, qui a étendu les moyens de l'autorité judiciaire et a permis l'ouverture d'une enquête à l'encontre de Jérôme Cahuzac au titre de blanchiment de fraude fiscale, ni de la procédure d'enquête judiciaire créée par la loi du 30 décembre 2009 de finances rectificative. Pour peu qu'on lui en donne les moyens, la justice française ne fait pas défaut

Ces arguments ne peuvent plus tenir devant les citoyens français, soucieux du respect des principes démocratiques. Ils ne tiennent plus devant les contribuables, qui voient le principe du consentement à l'impôt

aux citoyens, contribuables et justiciables, pouvons-nous prétendre à l'efficacité d'un dispositif permettant à l'administration fiscale de traiter certains dossiers, sans contradictoire, sans motivation des décisions

possible « une spécialisation du ministère public permettant d'accroître son action contre la très grande délinquance économique et financière, dont relève la fraude fiscale complexe ». De même, notre collègue de la commission des finances, que je salue, soulignait l'apport des techniques spéciales d'enquête dont bénéficient les services judiciaires dans les cas des fraudes les plus complexes. C'est bien dans ce cadre de collaborations que nous devons nous situer. Mes chers collègues, il est temps

je m'exprime ici alors que des semaines d'auditions ont eu lieu à l'Assemblée nationale. En ce moment même, les affaires dévoilées par la presse et les lanceurs d'alerte se succèdent ou sont en cours d'investigation. Chacune d'entre elles constitue un acte de résistance de la démocratie, ... Il faut conclure. ... mais en ébranlant l'opinion, elles agissent comme autant de crises de confiance, et c'est là le paradoxe. Allons-nous justifier le jusqu'à ce que la démocratie s'en trouve suffisamment affaiblie, ou bien allons-nous saisir l'occasion qui nous est donnée aujourd'hui de faire face aux responsabilités propres à notre fonction, en supprimant cette anomalie française qu'est le « verrou de Bercy »

allant vers plus de transparence, sans supprimer le verrou. Nous allons en égrener quelques-unes, bien avant le rapport de nos collègues de l'Assemblée nationale.

Je voudrais d'abord revenir sur le mécanisme de ce fameux verrou. Chaque année, l'administration conduit 1 million de contrôles sur pièces, mais surtout 50 000 contrôles fiscaux sur place. L'objectif du contrôle fiscal est triple recouvrer, sanctionner, dissuader. L'administration cherche donc à récupérer les droits et peut appliquer des pénalités allant de 40 % à 100 % selon les cas.

a limité aux cas les plus graves la possibilité de cumuler sanction administrative et sanction pénale. Sur les 50 000 contrôles fiscaux externes, 4 000 sont qualifiés de « répressifs À ce stade, nous n'en sommes pas encore au « verrou de Bercy », à proprement parler. Nous nous situons non pas au 139 rue de Bercy, mais dans les directions départementales des finances publiques,

ne peut déposer plainte que si elle y est autorisée par la CIF, ce qu'elle fait dans 90 % à 95 % des cas tant l'administration a intériorisé l'exigence de cette commission. Je préfère le dire avec solennité

la transparence est assurée par un certain nombre de rapports- rapport d'activité de la CIF, rapport au Parlement sur les remises et transactions, rapport du Comité du contentieux fiscal, douanier et des changes -, et ce sans compter les enquêtes menées régulièrement par la Cour des comptes. Ce n'est plus suffisant, vous l'avez dit, madame

Ces critères, réglés par circulaire, ont été en partie repris par le Conseil constitutionnel. Ce sont le montant des droits fraudés ; les manoeuvres du contribuable, qui constituent une circonstance aggravante ; les circonstances relatives à la personne même du fraudeur,

Gérald Darmanin a suggéré de faire entrer des parlementaires à la commission des infractions fiscales. Je ne pense pas que ce soit notre place ou notre mission, d'autant que le volume de travail de cette commission serait difficilement compatible avec notre agenda. En revanche, troisième proposition, pourrions envisager que des parlementaires, habilités à cet effet, contrôlent les 50 dossiers rejetés chaque année par la CIF, afin de comprendre les raisons pour lesquelles il a été décidé de ne pas les transmettre à la justice. Ces parlementaires pourraient également, par voie de sondage, examiner une partie des 3 000 dossiers non transmis par l'administration à la CIF. Bien entendu, ils devraient appartenir à tous les bords politiques, condition indispensable au rétablissement de la confiance. Un tel examen, qui permettrait de comprendre concrètement le fonctionnement du système, me paraîtrait plus efficace que l'audition annuelle de la CIF prévue par la loi de 2013. Quatrième proposition, les membres de la CIF désignés par les présidents des deux assemblées pourraient, plus logiquement, être proposés par le président et le rapporteur général des commissions des finances, afin d'assurer la pluralité.

d'un dossier ne sont pas suffisamment certaines, est-il pertinent de mettre sur la place publique la situation d'une personne ou d'une entreprise de bonne foi ? Je vois là une question de protection des personnes, mais aussi des intérêts économiques. j'en viens au monopole du dépôt des plaintes par l'administration. Cela répond à une logique très simple : l'État porte plainte parce que c'est lui la victime. comme le Sénat l'a déjà voté, peut-être faudra-t-il permettre à l'autorité judiciaire d'étendre une enquête existante à des faits de fraude fiscale connexes. Septième proposition, peut-être faudra-t-il aussi que la CIF puisse être saisie cette fois-ci

Monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, je suis très heureux d'intervenir devant vous aujourd'hui sur un sujet qui fait l'objet, cela vient d'être rappelé, de réflexions et de travaux approfondis, aussi bien au Sénat qu'à l'Assemblée nationale. En témoigne la mission

L'examen de cette proposition de loi issue du groupe socialiste et républicain m'offrira donc l'occasion, je l'espère, de dissiper un certain nombre de malentendus, qui semblent avoir été repris dès l'exposé des motifs du texte. Je

de le faire votre rapporteur, dont je salue l'objectivité, je m'attacherai donc à décrire les faits avec précision, tout en dessinant des pistes de réflexion pour pallier le manque de transparence dont- nous en convenons tous comme vous l'aurez constaté, le projet de loi relatif à la lutte contre la fraude que le Gouvernement a déposé sur le bureau du Sénat ne comporte pas de disposition sur le sujet.

De fait, le rejet du texte par votre commission des finances suffit, me semble-t-il, à démontrer que la démarche d'ouverture du Gouvernement a été entendue. Je ne surprendrai donc personne en annonçant que le Gouvernement n'est pas favorable à une suppression pure et simple du « verrou de Bercy ». En revanche, et ce sera l'objet de mon intervention, je souhaite que nous puissions remettre aux parlementaires les clefs de ce verrou, en sanctuarisant dans la loi les critères déclenchant des poursuites pénales en matière de fraude fiscale, tout en renforçant leurs pouvoirs de contrôle. rejoignons ainsi la position de votre rapporteur, qui propose lui aussi l'inscription de ces critères dans la loi et l'amélioration du contrôle sur la sélection de ces dossiers. J'ajoute, pour être complet, que le Gouvernement partage aussi pleinement les préoccupations du rapporteur en matière de préservation du secret fiscal. Ce dernier ne saurait être levé qu'en toute fin de procédure.

Est-ce si choquant ? Dans beaucoup d'autres domaines de l'action pénale, personne n'imaginerait que l'on puisse engager des poursuites sans une plainte de la victime. Or, en cas de fraude, c'est le Trésor qui est lésé ! C'est donc en tant que victime que l'administration fiscale porte plainte pour engager l'action pénale. En réalité, il y a derrière le sentiment que ce système est par trop verrouillé l'idée selon laquelle la fraude est non pas l'affaire d'experts, mais l'affaire de tous. C'est naturellement vrai. C'est d'ailleurs la le projet de loi relatif à la lutte contre la fraude généralise la publication des sanctions en matière pénale et permettra la publication des sanctions administratives. Pour autant, on voit mal comment les choses pourraient aller véritablement plus loin en la matière. Sans exigence de plainte préalable de l'administration, le juge judiciaire se retournera toujours vers l'administration fiscale pour caractériser la fraude et le dossier finira toujours par revenir chez l'expert Les finances publiques ne seront pas gagnantes à un changement de système, et la levée du « verrou » irait au-delà de notre objectif commun, qui est de sanctionner les fraudeurs et d'additionner aux sanctions administratives les sanctions pénales dans les cas les plus graves.

En réalité, non. Elle s'emploie surtout à vérifier que le dossier est suffisamment solide et étayé juridiquement pour que l'on mobilise l'autorité judiciaire, dont elle sait qu'elle a de nombreuses autres préoccupations et qu'il est peut-être inutile de l'engorger inutilement. Ce travail de filtre pose-t-il une difficulté ? Je ne le crois pas non plus, puisque la commission des infractions fiscales valide 85 à 95 % des propositions de plaintes selon les années. Par ailleurs,

qui oblige la commission à publier un rapport annuel et dispose qu'un débat sur son action doit avoir lieu chaque année devant les commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat. Le rapport prévu est élaboré chaque année et comporte des informations utiles. Le débat devant les commissions n'a jamais été organisé Faut-il pour autant laisser le système actuel en l'état, sans rien y changer ? Je ne le crois pas, et ce n'est pas la position du Gouvernement. S'il existe tant de fantasmes autour du « verrou de Bercy », cela signifie que des évolutions sont nécessaires. Je rejoins ici M. le rapporteur quant à la nécessité de réformer le dispositif afin d'y introduire plus de transparence sur les critères de transmission des dossiers à la CIF. Cela permettra de dissiper les fantasmes, parmi lesquels l'idée selon laquelle le ministre en charge du budget déciderait lui-même de la transmission des dossiers. Toutes les décisions de ne pas transmettre les dossiers à la CIF sont tracées et peuvent être auditées. Il y a donc sans doute de bonnes raisons de ne pas transmettre, soit que le dossier soit au contentieux devant le juge administratif, soit que la fraude ne soit, par exemple, pas suffisamment caractérisée. Aucune Aucune main invisible n'intervient pour protéger certains et en exposer d'autres. Votre rapporteur a souhaité, à ce titre, que des parlementaires habilités puissent mieux contrôler le travail de transmission de l'administration fiscale. Le Gouvernement est favorable à cette proposition. En réalité, comme Gérald Darmanin a eu l'occasion de le dire et de le proposer devant la mission d'information de l'Assemblée nationale, nous considérons que la loi devrait être plus claire sur les critères de définition des dossiers fiscaux donnant lieu à proposition de poursuite pénale, qu'il s'agisse du montant des droits fraudés, des agissements du contribuable ou encore du contexte du dossier. Je pense également que, en matière de présomption de fraude, c'est-à-dire lorsque la fraude n'est pas encore caractérisée, les instruments à disposition de l'administration n'étant pas suffisants, ou lorsque la démonstration de la fraude nécessite la mise en oeuvre de méthodes d'enquête beaucoup plus intrusives, le sas de la CIF n'est pas nécessaire. En effet, il s'agit non pas ici de rajouter une couche pénale aux sanctions déjà appliquées au niveau fiscal, mais de passer le témoin du contrôle fiscal à la police fiscale afin de poursuivre l'enquête. Le Gouvernement considère, en revanche, qu'une ligne rouge ne doit pas être dépassée : celle qui consisterait à remettre en cause le principe de plainte préalable de l'administration, en cas de connexité par exemple. C'est avant tout un sujet de coordination des procédures. Il faut veiller à ce que les choses soient faites dans l'ordre et à ne transmettre à la CIF que les dossiers les plus graves et pour lesquels l'application de sanctions pénales complémentaires aux sanctions administratives paraît justifiée.

dans laquelle, par exemple, un contribuable serait condamné pénalement pour fraude, mais verrait ses rappels et pénalités annulés devant le juge administratif. Deuxièmement, les procédures se multipliant, le nombre de dossiers dans lesquels sanctions pénales et sanctions administratives se cumuleront augmenterait nécessairement. Ce cumul de peines est, certes, admis par le Conseil constitutionnel, mais seulement dans les cas les plus graves. La nécessité d'un processus sélectif pour amener les dossiers au pénal est donc consubstantielle à ce principe. Elle s'imposera, quoi que l'on veuille, à toute évolution de notre procédure actuelle. Je note, d'ailleurs, que la procureur du Parquet national financier, le PNF, ne disait pas autre chose lorsqu'elle déclarait, en mai 2016, que « le rôle de filtre assuré par la CIF est une bonne chose, dans la mesure où il faut être pragmatique : la justice serait dans l'incapacité de traiter l'ensemble des plaintes En conclusion, vous l'aurez compris, le Gouvernement ne souhaite pas l'adoption de cette proposition de loi, tant la suppression complète et immédiate à la fois du monopole du dépôt des plaintes par l'administration fiscale et de la validation de la CIF aurait des conséquences sur l'engorgement de la justice ou l'efficacité dans le recouvrement des sommes dues et des pénalités. À vouloir tout judiciariser, nous risquons d'affaiblir l'efficacité de notre système répressif, ce qui serait contraire à l'objectif. La voie que nous vous proposons constitue une véritable amélioration de notre système. Elle consiste, comme je l'ai indiqué il y a un instant et comme l'a proposé votre rapporteur, à maintenir le « verrou », mais à vous en remettre les clefs, à vous, parlementaires, en définissant dans la loi les critères de transmission des dossiers et en renforçant vos moyens de contrôle, conformément au principe de la séparation des pouvoirs. Pour terminer, je veux vous répondre, madame la sénatrice Marie-Pierre

nous voulons d'abord saluer l'initiative de nos collègues du groupe socialiste et républicain de porter au débat la question du fameux « verrou de Bercy », sujet abordé à plusieurs reprises en commission des finances et dans l'hémicycle,

Chacun conviendra que, au lendemain du jugement rendu par la cour d'appel sur l'affaire Cahuzac- je suis désolé, mes chers collègues, de rappeler cet épisode terrible pour la République, mais l'actualité m'y amène -, ce débat sur le « verrou de Bercy » prend un tour particulier. de ses fonctions de ministre délégué au budget, Jérôme Cahuzac avait le privilège, par le mécanisme du « verrou de Bercy », de décider ou pas d'ester en justice contre lui-même. Convenez, mes chers collègues, que cette situation oscille quelque peu entre l'hallucinant et l'ubuesque Cette situation nourrit un sentiment de justice à deux vitesses chez nos concitoyens : les plus puissants semblent bénéficier d'une impunité inacceptable, il n'y a plus d'égalité devant l'impôt. Observons un instant les statistiques sur les 50 000 contrôles fiscaux réalisés chaque année, de 12 000 à 15 000, selon les années, mettent en évidence des fraudes caractérisées. Sur ce total, quelque 4 000 dossiers concernent un montant de fraude supérieur à 100 000 euros. Combien de gros fraudeurs finissent devant la justice ? C'est là que s'enclenche le « verrou de Bercy ». L'administration fiscale, qui fait un travail remarquable- rappelons-le sans cesse fait un premier tri entre ces 4 000 dossiers et détermine ceux qu'elle transmet à la commission des infractions fiscales, composée de magistrats du Conseil d'État, de la Cour des comptes et de la Cour de cassation. Puis, parmi les dossiers reçus, la CIF choisit à son tour ceux qu'elle transmet à la justice. En général, sur les 4 000 dossiers de gros fraudeurs, le fisc en transmet entre 900 et 1 000

que nos concitoyens s'indignent de cette situation quand, dans ce pays, on peut être condamné à deux mois de prison ferme pour avoir volé un paquet de pâtes alimentaires ? Non seulement le monopole de l'administration fiscale pour déclencher les poursuites en matière de fraude fiscale commise en bande organisée ou complexe est contre-productif, mais il heurte de front l'idéal de justice. On nous dit que l'actuel dispositif serait plus efficace lorsque, au cours des contrôles classiques, les agents identifient des indices de fraude fiscale qui pourraient laisser penser qu'ils sont en présence d'une fraude fiscale grave ou transnationale dans certains cas. Ils ne peuvent pas se satisfaire de simples indices. Ils doivent établir l'existence d'une présomption caractérisée qu'une infraction fiscale pour laquelle il existe un risque de dépérissement des preuves résulte des procédés figurant au livre des procédures fiscales. Or il n'est pas possible d'y parvenir sans mettre en oeuvre des moyens coercitifs dans le cadre d'investigations judiciaires qui, dans un État de droit, ne peuvent être autorisées que par une autorité judiciaire. C'est ainsi qu'il arrive que des indices ne soient ni traités ni transmis à la justice. Pour contrer l'action de l'administration, qui s'est révélée jusqu'à présent très efficace, les fraudeurs émiettent les intervenants en recourant à des prête-noms, des sociétés-écrans ou des entreprises fictives. Dans ces cas de fraudes très complexes, là encore, seules des enquêtes judiciaires permettraient de démonter les schémas de fraude. L'existence du « verrou de Bercy » n'est-elle pas aussi de nature à engendrer une confusion entre l'exécutif et le judiciaire ? Cette situation est-elle acceptable en démocratie ? Pourquoi les dossiers fiscaux très médiatisés de grands groupes transnationaux et de certains particuliers fortunés ne sont-ils pas parvenus à un juge d'instruction ? Personne ne nie ici que les agents du fisc aient une expertise incomparable. Mais les magistrats disposent de techniques spéciales d'enquête indispensables dans les affaires impliquant la criminalité organisée ou faisant intervenir sociétés-écrans et logiciels comptables frauduleux. Croit-on vraiment que les grands groupes cesseront de tricher tant qu'aucune condamnation pénale ne les dissuadera, par exemple, de manipuler les prix de transfert ? Les intermédiaires arrêteront-ils de conseiller et de protéger les fraudeurs tant que l'impunité leur sera garantie ? Mes chers collègues, ce « verrou de Bercy » n'a plus aucune légitimité depuis la création, en 2013, du Parquet national financier, le PNF, qui a justement compétence sur les infractions fiscales graves.

Lors de son audition par la commission spéciale de l'Assemblée nationale, celle-ci a déclaré que « le verrou de Bercy bloque toute la chaîne pénale », qu'il « empêche la variété des poursuites et constitue un obstacle juridique » et « un handicap sur le plan pratique ». Les procureurs, censés diriger l'action publique, en sont réduits à attendre de voir arriver une petite partie du spectre de la fraude fiscale que Bercy souhaite leur transmettre. La liberté d'action du PNF est mise à mal par le « verrou de Bercy ». La phase administrative, la sélection et le choix des affaires qui doivent faire l'objet de poursuites échappent totalement au Parquet national financier, qui a transmis, l'an dernier, 77 signalements de suspicion de fraude fiscale à Bercy, mais n'a aucun moyen de savoir à l'heure actuelle comment ces cas graves ont été ou seront traités. Un parlementaire compromis ne pourrait pas être jugé pour fraude fiscale sans une plainte de Bercy. Cela pose évidemment et de manière très concrète la question des moyens financiers, techniques et humains de la justice. Il faut conclure, mon cher collègue. La réduction de la dépense publique a aussi des conséquences pour les magistrats.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, monsieur le vice-président de la commission des finances, monsieur le rapporteur, mes chers collègues,

diagnostiqué cette anomalie, dont plusieurs personnes auditionnées avaient soutenu la suppression.

Le groupe Union Centriste n'est pas favorable, dans sa majorité, à la suppression pure et simple du « verrou », qu'à titre personnel, je voterai. Toutefois, nous avons proposé un amendement d'assouplissement. Puisque

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, monsieur le vice-président de la commission, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, chaque année, la fraude fiscale représente une perte de 60 à 80 milliards d'euros pour le budget de la France. donnent le vertige, parce qu'elles représentent environ 15 % du budget de l'État. Au plan international comme au plan national, grâce aux lanceurs d'alerte, aux médias, aux ONG, qui ont alerté les citoyens et poussé les gouvernements à légiférer, des avancées incontestables ont été opérées ces dernières années.

texte est une fin en soi, parce qu'il abroge un système inacceptable sur les principes, mais il n'est pas un aboutissement, car d'autres mesures sont indispensables pour mettre sur pied un système alternatif pleinement efficace. Qu'appelle-t-on « le verrou de Bercy » Aujourd'hui, même si c'est toute la société qui est spoliée par les fraudeurs, la seule entité en droit de porter plainte pour fraude fiscale est le ministère des comptes publics. Nous sommes les seuls dans le monde à appliquer une telle règle, au mépris du principe le plus fondamental de la démocratie : la séparation des pouvoirs.

Supprimer le « verrou de Bercy » est la seule manière de lutter contre cette impression de collusion des élites qui s'assemblent pour reporter la charge fiscale sur les citoyens. En effet, aller devant le juge, écoper d'une sanction pénale a une connotation morale essentielle et dissuasive. Face aux divers scandales, qui se répètent, les citoyens, qui, eux, ne peuvent pas « s'évader », nous interpellent et nous regardent. Le doute devant le manque de justice fiscale est présent chez tous les contribuables qui s'acquittent de leurs impôts et qui ne comprennent pas que certains puissent réaliser des « montages exotiques » pour optimiser leur fiscalité ou cacher une partie de leurs revenus ou patrimoines. C'est aussi au nom de la concurrence déloyale que cette fraude doit être pénalement punie. Actuellement, la droiture est une faiblesse qui dessert la compétitivité des entreprises vertueuses, face à celles qui ne jouent pas le jeu. D'ailleurs, c'est sous cet angle de la concurrence déloyale que la commissaire européenne à la concurrence, Mme Vestager, a jugé que le régime fiscal dont bénéficie, par exemple, Apple en Irlande est assimilable à des aides publiques indues

On nous parle souvent de mutualisation, de rationalisation. Pour le coup, dans le système actuel, on a empilé les dispositifs sans les articuler : la commission des infractions fiscales, qui, comme cela a été dit, sert de filtre totalement opaque entre le ministère des finances et le parquet, analyse un quart des dossiers dits « répressifs », autrement 10 % des mêmes dossiers sont suivis par la Brigade nationale de répression de la délinquance fiscale, la BNRDF. Il est question d'ajouter une nouvelle police fiscale, dont l'articulation avec la BNRDF est floue. Si l'on ajoute à cela que la police des douanes traite principalement de fraudes à la TVA, on réalise que le système est particulièrement complexe

4 000 fraudes d'une gravité particulière ... Il est quand même paradoxal de qualifier d'efficace un système qui ne fait pas baisser le nombre de fraudes. Il est tout aussi paradoxal, et même intolérable, de considérer comme efficace permet de recouvrer que 5 à 10 % du montant total estimé de la fraude. Pour ma part, je n'appelle pas cela un système efficace, d'autant que ce système est porteur d'effets pervers, l'administration intégrant en amont les règles de filtrage.

aboutissant à des peines pénales. Il faut lever le doute sur une possible sélection qui tiendrait compte du CV du contribuable plus que de l'infraction. On nous oppose aussi souvent que les juges n'ont pas le temps, ne sont pas formés, ne s'intéressent pas à ces affaires. Il est exact que les enquêtes sont souvent limitées et ne vont pas plus loin que les dossiers transmis par les contrôleurs des impôts. Il est exact que de nombreux juges, dans les petits tribunaux notamment, sont

d'autant que le Parquet national financier est doté de moyens insuffisants et que, dans le même temps, les effectifs des pôles économiques et financiers des parquets des tribunaux de grande instance diminuent. Le système qui s'est construit autour du « verrou de Bercy » est à bout de souffle. Les lois précédentes ont permis de tracer les contours d'un système alternatif, fondé sur une coopération renforcée entre juges et administration fiscale,

Le Conseil constitutionnel a jugé qu'une double sanction pouvait s'appliquer pour les cas présentant un caractère exemplaire ou grave de par l'importance des montants en cause ou la complexité du dispositif de fraude mis en oeuvre. Ces définitions devront nous permettre d'automatiser la transmission de ces cas graves ou complexes à la justice pénale.

insiste sur les moyens humains nécessaires aux enquêtes judiciaires menées par la BNRDF. Il est question, dans le projet de loi de M. Darmanin, de la création d'un autre service, dont on comprend mal le lien avec la BNRDF, et d'une quarantaine d'agents en redéploiement

On affiche des sanctions de plus en plus sévères- selon le projet de loi Darmanin, il serait question d'aller plus loin encore -, mais ces peines sont rarement appliquées : beaucoup de communication, peu d'efficacité Au Royaume-Uni, en Italie, des peines de prison ferme sont bien plus souvent prononcées. En outre, le juge peut avoir recours aux travaux d'intérêt général, peine qui présente un caractère d'exemplarité très fort. Il s'agit d'une première piste de réflexion

L'inscription au casier judiciaire est rarement retenue. Ne pourrait-elle l'être beaucoup plus systématiquement ? À l'égard de la petite délinquance, on n'a pas ce genre de pudeur ... Enfin, il faut clarifier la distance entre fraude et optimisation fiscale, car c'est dans cette zone grise que tout se passe.

Je vais le dire assez clairement pour qu'il n'y ait pas de suspense : une suppression sèche de ce dispositif, c'est-à-dire sans réfléchir à un mécanisme de substitution ou à d'éventuelles améliorations, me semble, pour plusieurs

On ne légifère pas non plus sous la pression médiatique ou sous la pression des effets de mode, encore moins au Sénat. Mes chers collègues, la vocation de la Haute Assemblée de se prémunir contre ce qui se passe malheureusement trop souvent à l'Assemblée nationale. À force de subir la pression médiatique, les effets de mode, on finit par regretter d'avoir élaboré des lois totalement

et d'obtenir une restitution la plus rapide possible des sommes non recouvrées. L'administration fiscale me semble donc dans son rôle lorsqu'elle recourt à la transaction pour récupérer efficacement les sommes soustraites à la collectivité. Là est l'intérêt général. J'ajoute que ceux qui dénoncent l'engorgement des tribunaux sont ceux-là mêmes qui poussent à une surpénalisation. Mes chers collègues- je m'adresse principalement à ceux qui veulent vraiment lutter contre la fraude fiscale -, si vous voulez enterrer un dossier,

de le laisser pourrir. Par ailleurs, les procédures de règlement amiable des différends en matière fiscale me semblent aller dans le sens de l'avenir et de la modernité.

Nous partageons la volonté de changement des auteurs de ce texte, mais nous estimons que cette proposition de loi est à la fois trop brutale et prématurée, raison pour laquelle le groupe Les Indépendants - République

la question que pose le « verrou de Bercy » est celle de la séparation des pouvoirs et de la transparence dans les relations entre administration fiscale et autorité judiciaire.

En effet, en vertu de l'article L. 228 du livre des procédures fiscales, « les plaintes tendant à l'application de sanctions pénales en matière d'impôts directs, de taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes sur le chiffre d'affaires, de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière et de droits de timbre sont déposées par l'administration sur avis conforme de la commission des infractions fiscales », et ce sous peine d'irrecevabilité. Toujours selon le même article, « la commission examine les affaires qui lui sont soumises par le ministre chargé du budget. Le contribuable est avisé de la saisine de la commission qui l'invite à lui communiquer, dans un délai de trente jours, les informations qu'il jugerait nécessaires. L'administration fiscale possède donc le monopole du déclenchement de poursuites pénales en matière de fraude fiscale. Ce privilège légal remonte aux années 1920, à une époque où l'État souhaitait recouvrer plus efficacement les impôts. Il faut le reconnaître, l'État, le « plus froid de tous les monstres froids », comme l'a appelé Nietzsche, se préoccupe plus souvent d'efficacité que d'éthique. Mais cette particularité a-t-elle encore une raison d'être aujourd'hui ? Le « verrou de Bercy » est un sujet bien connu au Sénat. Nous en avons débattu à maintes reprises, ces dernières années. Il est déjà arrivé à notre assemblée de voter sa suppression ou, à tout le moins, son assouplissement.

prévoyant la levée du « verrou de Bercy » pour fraude fiscale associée à d'autres activités criminelles ou délictuelles avait été adopté. Je rappellerai également que le groupe du excellent collègue Pierre-Yves Collombat, avait proposé de confier l'initiative de poursuites au procureur de la République financier sur avis simple de la commission des infractions fiscales. infractions fiscales. S'il avait reconnu la légitimité du débat, Michel Sapin avait néanmoins émis un avis défavorable, considérant que l'efficacité du dispositif devait primer sur les considérations éthiques.

un transfert brutal à l'autorité judiciaire sans dispositif transitoire- engorgement, perte d'expertise, de confidentialité ... Toutefois, les arguments en faveur d'une plus grande transparence, notamment s'agissant des critères de sélection des dossiers transmis par la CIF au juge pénal- montant concerné par la fraude, agissements du contribuable, circonstances personnelles -gardent toute leur pertinence. Le manque de données sur le nombre de dossiers traités, l'ampleur des affaires celle des transactions contribuent à la crispation des positions sur ce débat, ce qui n'est ni sain ni acceptable. Il faut néanmoins souligner les progrès accomplis ces dernières années. Même s'il reste du chemin à parcourir pour en finir avec la fraude, un changement de culture, comme le rappelle l'exposé des motifs de la proposition de loi, s'est opéré et la lutte contre l'évasion fiscale a gagné en efficacité. De nouveaux outils ont été créés. Je pense à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique et au Parquet national financier. Après l'affaire Cahuzac, la Haute Autorité a rendu publics des manquements ayant entraîné la démission de deux anciens ministres. Chargé des affaires les plus complexes, le Parquet national financier a obtenu quelques condamnations fortes et symboliques. La loi Sapin II de 2016 a notamment accordé un statut aux lanceurs d'alerte, créé l'Agence française anticorruption et introduit l'infraction pour corruption d'agent public étranger. Enfin, le guichet pour les fraudeurs repentis, ouvert entre 2013 et 2017, a permis de régulariser quelque 32 milliards d'euros d'avoirs et de recouvrer près de 8 milliards d'euros. La présente proposition de loi permettrait, si elle était adoptée, d'approfondir logiquement ce changement culturel. C'est la raison pour laquelle les membres du groupe du RDSE sont, dans leur très grande majorité- à une exception près

droit commun. L'administration opérant un filtre, ce manque de transparence est critiqué. D'aucuns pensent que des affaires de fraude fiscale sont ainsi étouffées. En réalité,

Dans sa décision du 22 juillet 2016, le Conseil constitutionnel estime que ce mécanisme ne porte pas « une atteinte disproportionnée au principe selon lequel le procureur de la République exerce librement [ ...] l'action publique ». Une fois la plainte déposée, le parquet a « la faculté de décider librement de l'opportunité d'engager des poursuites. » Par ailleurs, le Conseil constitutionnel juge que l'administration fiscale est la mieux placée pour estimer le préjudice qui lui est causé par la fraude fiscale et qu'ainsi « l'absence de mise en mouvement de l'action publique ne constitue pas un trouble substantiel à l'ordre public. Enfin, le « verrou de Bercy » s'inscrit, selon le Conseil constitutionnel, « dans le respect d'une politique pénale déterminée par le Gouvernement ». Par ailleurs, ce dispositif est encadré par une autorité administrative indépendante- la commission des infractions fiscales composée de membres du Conseil d'État, de conseillers de la Cour des comptes, de magistrats de la Cour de cassation et de personnalités qualifiées nommées par les présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale. C'est elle qui décide du dépôt de plainte ou non. Dans les faits, 90 % des dossiers qui lui sont transmis font l'objet d'une plainte. En amont de cette commission, l'administration fiscale effectue un travail de contrôle : chaque année, elle opère 1 million de contrôles sur les pièces transmises pour la déclaration d'impôt et 50 000 contrôles fiscaux. Elle réalise un travail d'investigation très pointu qu'un magistrat pénal ne pourrait effectuer aussi rapidement et facilement, facilement, ne disposant pas de l'expertise technique de Bercy. Il aurait, de toute façon, besoin des services de l'administration pour être éclairé. En outre, le secret fiscal est parfaitement préservé par Bercy, ce qui n'est, hélas !, pas toujours le cas du secret de l'instruction. Nous avons pu constater à plusieurs reprises que, de manière très sibylline,

année 4 à 5 milliards d'euros de recettes pour l'État, à moins d'embaucher des centaines de magistrats pour examiner les 16 000 manquements délibérés et les 4 000 dossiers répressifs constatés en matière de fraude fiscale.

nécessaires, nous n'en disconvenons pas. Ainsi, les critères de sélection des dossiers par Bercy et par la commission des infractions fiscales, aujourd'hui définis par une circulaire, devraient être redéfinis par la loi.

Des amendements allant dans ce sens seront d'ailleurs déposés dans le cadre du projet de loi relatif à la lutte contre la fraude qui sera examiné prochainement par le Sénat, première chambre saisie de ce texte. Dans l'attente de l'examen de ce projet de loi, et pour toutes les raisons que je viens d'évoquer, le groupe Les Républicains n'adoptera pas cette proposition de loi, conformément à la position de la commission des finances et de son rapporteur, Jérôme Bascher, que je tiens à

Monsieur le président,

des temps de réflexion et de débats, même si nous avons parfois le sentiment d'être répétitifs, à l'efficacité de la collecte de l'impôt. À cet égard, je veux remercier Mme Marie-Pierre de la Gontrie d'avoir déposé cette

Nous avons le choix entre deux extrémités également condamnables : faire de Bercy et de l'administration le « cercle des dossiers disparus », ce qui donnerait le sentiment d'une obscurité coupable, coupable, ou accepter le pilori en place de Grève, avant qu'il y ait eu instruction et,, condamnation, ce qui est malheureusement souvent le cas

Sans doute avait-il eu la volonté de faire en sorte que ce secret soit maintenu, pour préserver l'égalité des citoyens et ne pas les exposer à la pression de Bercy,

à une solution définitive. Il serait malheureux d'abandonner une procédure qui rend implicitement au sérieux, à la responsabilité, au professionnalisme, mais aussi- et ce n'est pas sans importance -à la discrétion de l'administration des impôts, laquelle est assurément un facteur de cohésion et de respect de l'État pour l'ensemble des citoyens,

939 condamnations, dont 430 définitives ; 360 peines de prison, dont seulement 68 fermes, mais, pour l'essentiel d'entre elles, faisant l'objet d'aménagements ; et et 131 peines d'amende, dont 121 fermes, pour un montant moyen de 14 000 euros, ce qui est évidemment bien éloigné de la moyenne de 453 000 euros que j'évoquais voilà un instant. Des questions ont été posées à propos de la police fiscale prévue dans le cadre du projet de loi relatif à la lutte contre la fraude, qui sera bientôt présenté devant votre assemblée. Je veux le rappeler, la procédure d'enquête fiscale a été créée pour permettre d'asseoir l'impôt. À cette fin, les officiers fiscaux judiciaires ont été dotés de prérogatives de police judiciaire permettant auditions, gardes à vue, perquisitions, saisies judiciaires et écoutes. Ainsi, 83 % des plaintes déposées par la DGFiP concernent la fraude fiscale sophistiquée, qui a recours à des montages opaques et au blanchiment, et non pas le crime organisé. Ces fraudes doivent mobiliser une expertise avant tout fiscale. Les résultats obtenus par la Brigade nationale de répression de la délinquance fiscale, évoquée précédemment, sont sont contrastés, puisque 496 plaintes ont été déposées par la DGFiP depuis 2010 ; 124 dossiers fiscalisés par la DGFiP ont permis 209 millions d'euros d'impôts et de pénalités mis en recouvrement 62 décisions de justice sont intervenues, dont 12 classements sans suite ; 260 plaintes restent en cours, auxquelles il faut ajouter les 69 affaires de blanchiment de fraude fiscale, dans le cadre de l'affaire dite des « Panama Papers ». Au vu des capacités de traitement de la Brigade, soit environ 50 affaires par an, il faudrait six ans pour que le stock d'affaires en cours soit purgé. La création d'une police fiscale à Bercy est donc prévue à l'article 1 du projet de loi relatif à la lutte contre la fraude.

de privilégier une approche fiscale pour accélérer les rentrées budgétaires et, surtout, de densifier la coopération entre Bercy et la justice, en plaçant ce nouveau service sous l'autorité directe d'un magistrat de l'ordre judiciaire et, ainsi, d'avoir plus d'efficacité.

lui permettre de s'équiper des outils nécessaires, notamment en termes de collecte et d'analyse de données, et de mettre ainsi à profit la dématérialisation croissante, pour ne pas dire presque totale, des déclarations et des informations faisant l'objet de traitements et d'enquêtes, afin d'être plus efficace dans la recherche de la fraude.

pour obtenir les informations nécessaires, notamment celles qui permettent d'auditer et de tracer les décisions de la CIF ne donnant pas lieu à une transmission devant la justice. À cet

défriché le sujet. La discussion générale est close. La commission n'ayant pas élaboré de texte, nous passons à la discussion des articles de la proposition de loi initiale.

Le scrutin est ouvert.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

d'autre part, lorsque les faits ont été commis en bande organisée ou par le recours à diverses manoeuvres. Il vise en outre à ouvrir, sous le contrôle du parquet, une possibilité de transaction pénale pour les faits de fraude fiscale complexe commis dans les circonstances susvisées. Il s'agit donc d'un aménagement préfigurant tous ceux que vous suggérerez ou validerez dans le cadre du projet de loi qui nous sera soumis dans quelques semaines.

S'agissant de l'égalité entre les citoyens, au nom de quoi introduirait-on une procédure spéciale pour certains cas de fraude fiscale ? Toutes les affaires graves doivent aller devant le juge pénal, qu'elles relèvent ou non des conditions fixées par cet amendement. C'est justement l'avantage de la procédure actuelle, qui permet l'application de critères homogènes grâce au contrôle de la CIF. Il convient également de réfléchir au périmètre du mécanisme prévu par l'amendement. Les cas de fraude fiscale aggravée sont ceux qui justifient le plus le renvoi devant l'autorité judiciaire, mais ce sont aussi ceux ceux pour lesquels la compétence technique de l'administration est essentielle. Cela ne s'oppose en rien au dépôt de plainte. Certes, il manque à l'administration des moyens spéciaux pour mener l'enquête,

S'agissant de la première partie de l'amendement, c'est précisément lors des débats portant sur ce point que l'Assemblée nationale a décidé de constituer une mission d'information.

Un certain nombre de choses ont été faites au cours du précédent quinquennat, notamment la création du Parquet national financier- cela a été rappelé. Des dispositifs ont été mis en place- ils sont désormais opérationnels

et faire cesser cette logique qui n'est pas du tout dissuasive. Or il faut que nous entrions dans une logique dissuasive ! Oui, nous serons présents lors de la discussion du projet de loi Darmanin. Vous nous trouverez ici même, avec des propositions. Mais il eût été possible, et souhaitable, que le Parlement prenne ses responsabilités aujourd'hui,

de Mme Goulet, qui consiste à développer le recours à la transaction pénale en cas de refus de la solution transactionnelle durant la phase administrative, constitue un compromis intéressant, et

dans l'hypothèse d'instructions connexes. Ce n'est quand même pas la mer à boire, d'autant plus que l'article 1 de cette proposition de loi a déjà été rejeté par le Sénat et que le texte n'a aucune espèce de chance d'arriver jusqu'à l'Assemblée nationale, puisque nos collègues du groupe Les Républicains ont demandé un deuxième

Le scrutin est ouvert.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

Le scrutin est ouvert.

Monsieur le président, si vous

mon intervention se fonde sur l'article 36 du règlement. Le 7 mars dernier se tenait ici même une discussion houleuse sur la proposition de loi que nous allons de nouveau étudier ce soir.

Face à ce coup de force sans précédent et antidémocratique, nous avions suspendu l'examen de notre proposition de loi. Depuis, les retraités agricoles et des élus de toute la France se sont mobilisés et nous ont fait parvenir plus de 8 000 pétitions demandant expressément à votre gouvernement de revenir sur sa position et d'accepter de revaloriser les pensions agricoles sans attendre. Ces plus de 8 000 pétitions, je vais vous les remettre, madame la ministre, monsieur le secrétaire d'État. Elles seront entre vos mains, tout comme le devenir des retraités agricoles, dont certains, ce soir, sont de nouveau en tribune, aux côtés d'André Chassaigne, initiateur de cette proposition de loi à l'Assemblée nationale. Par ce rappel au règlement, je vous demande, madame la ministre, monsieur le secrétaire d'État, d'une part, si le gouvernement que vous représentez est prêt à faire un pas vers la démocratie en acceptant le débat sans avoir recours au vote bloqué, part, s'il est enclin à revoir son jugement sur le sort des pensions agricoles. À l'heure où le Sénat rassemblé

Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, mon intervention, comme celle de ma collègue Cécile Cukierman, se fonde sur l'article 36 du règlement. Ce matin, nous avons eu un débat, en commission des affaires sociales, sur cette proposition président, rapporteur, commissaire, a pu y exprimer son point de vue. Ce dialogue contrasté, parfois contradictoire, est nécessaire, utile, sain, et fait partie de l'exercice parlementaire. Je pense sincèrement qu'en politique, la confrontation est salutaire, et je ne suis pas seule à le penser : cette position est partagée,

pour les collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise agricole, les conjoints participant aux travaux et les aides familiaux, et ce seulement, mes chers collègues, en 2020 ! Quel mépris ! Il faut encore attendre Quelle générosité, mais surtout quel mépris pour le monde agricole ! Il en va de même avec votre amendement sur les travailleurs inaptes. Quel mépris, aussi, pour l'initiative parlementaire et pour l'esprit de consensus dont ont fait preuve les membres de la Haute Assemblée ! À l'aube de la réforme constitutionnelle voulue par le chef de l'État afin d'améliorer l'efficacité du travail parlementaire, vous avouerez que c'est la marque d'une cruelle ironie. En quoi maltraiter l'initiative parlementaire peut-il être gage d'efficacité, d'autant que, vous le savez bien, l'adoption de ces amendements entraînerait la fin de cette proposition de loi, une navette ne pouvant aboutir

Je tiens, par ce rappel au règlement, à vous faire part, madame la ministre, monsieur le secrétaire d'État, du soutien que notre proposition de loi a recueilli auprès de nombreux élus locaux. Car, au-delà des premiers concernés, les retraités eux-mêmes, la discussion et l'adoption de ce texte répondraient à plusieurs enjeux essentiels pour nos territoires. Il est urgent de faire bénéficier chaque agriculteur d'une pension décente au moment où il cesse son activité, pour plus de justice sociale d'abord, mais aussi parce que le niveau des retraites agricoles a un impact sur notre modèle agricole. Si nous voulons une agriculture avec des agriculteurs, si nous voulons résister aux phénomènes de financiarisation de l'activité agricole et d'accaparement des terres, il est impératif de permettre des départs anticipés des départs anticipés et des rachats d'exploitations à un coût acceptable, rendant possible l'installation de jeunes agriculteurs et la préservation d'un modèle d'agriculture à taille humaine. Répondre à la détresse des retraités agricoles, c'est faire le choix de maintenir une diversité des agricultures, des produits, des terroirs. C'est refuser une agriculture standardisée aux mains des firmes financières, avec des acteurs économiques capitalistiques en lieu et place des agriculteurs et de leur statut.

vous est donné de ce rappel au règlement,

de la Constitution, sur l'ensemble de la proposition de loi, modifiée par l'amendement n° 3, qu'il avait déposé. Pour la clarté de nos débats et afin de répondre d'ores et déjà aux différentes interrogations et d'éviter tout risque d'incompréhension, je me permets de vous apporter quelques précisions sur le déroulement de nos travaux. Dans le cadre de la procédure du vote unique, les sénateurs conservent la possibilité de prendre la parole sur tous les articles du texte, et les auteurs des amendements conservent naturellement leur droit de présentation. En conséquence, à chaque article, les sénateurs inscrits pour une prise de parole sur l'article disposent, en vertu de notre règlement, de deux minutes À l'issue de ces prises de parole et de la présentation des amendements, nous passerons aux explications de vote et au vote unique sur les articles, sur les amendements retenus et sur l'ensemble de la proposition de loi.

les conjoints collaborateurs sont ceux qui perçoivent les pensions les plus faibles, de l'ordre de 597 euros par mois. La pension majorée de référence est un minimum de pension de retraite de base spécifique au régime des non-salariés agricoles qui permet précisément de relever les pensions les plus faibles à un minimum variable selon la durée de cotisation. Le montant perçu par les conjoints qui travaillent sur l'exploitation est inférieur à celui qui est perçu par le chef d'exploitation. De fait, il reste à un niveau particulièrement bas : 546,17 euros par mois pour une carrière complète en tant que collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole ou aide familial. amendement vise donc à augmenter le minimum de pension des conjoints de 5 %. L'augmentation interviendra dès le 1 janvier 2020. Cette mesure de justice permettra d'améliorer la retraite de près de 160 000 personnes.

cet amendement représenterait, pour les intéressés, une augmentation de 27 euros par mois maximum, pour les assurés collaborateurs ayant effectué l'intégralité de leur carrière au sein du régime des non-salariés agricoles.

30 %. D'après les estimations fournies par le Gouvernement, le coût d'une telle mesure s'élèverait à 30 millions d'euros par an en moyenne, contre- je le signale -400 millions d'euros pour l'ensemble de la proposition de loi en débat aujourd'hui. L'amendement n° 5, quant à lui, à lui, vise à assouplir les conditions d'éligibilité aux points gratuits du régime complémentaire obligatoire des chefs d'exploitation pour les pensionnés actuels reconnus travailleurs inaptes ou handicapés ayant liquidé leur pension depuis 1997 en levant la condition du taux plein pour bénéficier de points gratuits et en alignant les règles. La commission des affaires sociales

monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, à la lecture de cette proposition de loi, je ne peux qu'approuver le principe d'une revalorisation des petites retraites agricoles, tout en émettant quelles remarques. En effet, la revalorisation des petites retraites en agriculture est un problème récurrent, que nous ne sommes jamais parvenus à endiguer, même si le passage de 75 % à 85 % du SMIC est une avancée.

elle-même due à la faiblesse des revenus. Aussi, cette revalorisation est une attente forte des anciens agriculteurs, qui voient tous les jours leur pouvoir d'achat diminuer. Et les décisions du Gouvernement, comme la hausse de la CSG et des carburants, n'ont fait qu'aggraver cette situation. Je formulerai deux remarques. La première concerne le mode de financement de cette revalorisation, qui représente environ 400 millions d'euros. la présente proposition de loi, il est prévu qu'elle soit compensée par l'augmentation de la taxe sur les transactions financières, portée de 0,3 % à 0,4 %. Il ne faudrait pas que cette compensation devienne très vite un leurre et que cela se termine par une énième augmentation de la cotisation des actifs à la retraite complémentaire obligatoire, ou RCO. En effet, la RCO, qui est de l'ordre de 760 millions d'euros, est aujourd'hui financée par la contribution des actifs, à hauteur de 470 millions d'euros, le reste étant compensé par des taxes diverses. Depuis 2014, la RCO des actifs n'a cessé d'augmenter, en passant de 3 % à 3,5 %, puis 4 %, pour atteindre l'objectif d'une retraite à 75 % du SMIC. Si ma crainte se révèle fondée, cela se traduira par un quasi-doublement de la cotisation à la RCO des agriculteurs actifs. Ce n'est absolument pas acceptable. Ma seconde remarque s'inscrit dans une réflexion plus globale sur la situation de nos agriculteurs. Comme les petites retraites résultent de petits revenus, leurs faibles montants résident dans la difficulté pour les agriculteurs de bénéficier de prix de vente de leurs produits suffisamment élevés. Une des raisons, largement connue, est la pression qu'exercent les enseignes des grandes surfaces pour faire baisser les prix depuis des décennies. Alors, au lieu d'augmenter la taxe sur les transactions financières pour compenser le coût de la revalorisation, ne faudrait-il pas augmenter la fiscalité des grandes et moyennes surfaces, la taxe sur les surfaces commerciales, ou TASCOM, et affecter ce produit à la revalorisation des retraites ? C'est le sens de la proposition de loi que j'ai aussi déposée sur la revalorisation des retraites agricoles. Il faut conclure, mon cher collègue. Cela permettrait enfin un juste retour du fruit du travail du laboureur et de ses enfants Certes, la terre n'est pas obligatoirement un trésor. Mais les grandes enseignes, comme Leclerc, Auchan et d'autres encore, s'en sont fait un sur le dos des paysans

par la retraite de misère de nos parents et grands-parents. Cela nous ramène aujourd'hui au sort de nombreux retraités agricoles. Aussi, cette proposition de loi constitue un appel à la dignité pour nos agriculteurs. Elle est un appel à la justice pour nos territoires ruraux.

Cette proposition de loi a déjà fait l'objet d'un vote à l'unanimité à l'Assemblée nationale. Et pour cause ! Elle répond à des situations de détresse de nos anciens chefs d'exploitation agricole, désormais à la retraite, dont un sur trois touche une pension de moins de 350 euros par mois, et dont le niveau moyen est le plus faible des régimes. La proposition de loi demande ainsi d'offrir un minimum que tout un chacun est en droit d'attendre après une vie de travail sans avoir jamais sollicité d'aides sociales diverses, sans avoir jamais sollicité la solidarité nationale, alors que les enfants accompagnent bien souvent leurs parents et leurs grands-parents en fin de Le désarroi dans lequel vivent certains de nos retraités mérite une action. Il ne peut pas attendre d'être traité dans le cadre d'un projet de réforme globale des régimes de retraite qui en est toujours au stade de l'annonce. Cette préoccupation a été celle de gouvernements successifs depuis 2002, notamment en 2011, où le régime de retraite a été élargi. Mais 75 % du SMIC, c'est assurément insuffisant ; 85 %, c'est un minimum vital Georges Pompidou, Président de la République, qui connaissait bien la ruralité du Cantal et la rudesse de la vie des agriculteurs, témoignait ainsi : « Mon père et ma mère appartenaient profondément à la race française, dure au travail, économe, croyant au mérite, aux vertus de l'esprit, aux qualités du coeur. Je n'ai pas eu une enfance gâtée. Mais, si loin que je remonte, je n'ai reçu que des leçons de droiture, d'honnêteté et de travail. Il en reste toujours quelque chose.

l'article. Madame la ministre, vous persistez ! Vous persistez à considérer que cette proposition de loi est prématurée. Nous, nous persistons à dire qu'il y a urgence sociale.

nous parlons pas le même langage. Vous nous parlez d'équilibre des comptes ; nous parlons de justice sociale et de nécessaire solidarité. On nous dit que cette proposition de loi est prématurée. Nous, nous disons qu'il y a une urgence sociale et que, par exemple, la réforme de l'impôt de solidarité sur la fortune n'était aucunement une urgence sociale ou une nécessité

envisagé de mettre à contribution le monde de la finance. En quoi cela peut-il gêner de prélever un centime d'euro pour l'achat d'une action de dix euros ? Vous nous parlez de chiffres et d'équilibre des comptes. Des chiffres, en voici, madame la ministre retraite de monsieur, non-salarié agricole dans le département de l'Aude, 646 euros ; retraite de madame, non-salariée agricole dans le département de l'Aude, 321 euros total, pour ce couple, 967 euros de retraite par mois ! Ne pensez-vous pas qu'un effort supplémentaire puisse être fait et qu'il y a urgence en la matière ? Voilà la situation difficile, pour ne pas dire précaire, dans laquelle se trouvent les anciens travailleurs de la terre après des décennies de dur labeur. Ils ne demandent donc que reconnaissance et justice sociale. Au cette demande urgente concerne en priorité non pas les grands propriétaires terriens, mais les petits paysans de métropole et d'outre-mer, ceux qui, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, ont fait passer l'agriculture autarcique à une agriculture de production. Ils ont droit à notre reconnaissance

en cette période difficile que traversent le monde agricole et le monde de l'économie rurale, lorsque je songe à ceux qui ont construit la richesse de notre pays pendant des décennies, J'ai honte de voir que l'on ne reconnaît pas la qualité de leur travail, la qualité de la production, la sécurité qu'ils apportent à nos besoins alimentaires au quotidien.

collègues, les pensions de retraite sont un enjeu vital pour nos agriculteurs. C'est d'autant plus vrai dans nos territoires ultramarins, à plus d'un titre. En Martinique, notre agriculture est soumise à des contraintes insulaires- ou à la dépendance économique vis-à-vis de certains produits d'importation -, climatiques, sanitaires, par exemple, la pression parasitaire, et à des possibilités réduites d'économies d'échelle, du fait de la prédominance des petites exploitations, du coût de la main-d'oeuvre et du prix élevé du foncier qui augmentent les coûts de production. Les coûts post-récoltes sont également élevés, en raison de la faible taille et de l'isolement des opérateurs concernés, rendant certains produits issus de l'agriculture locale peu compétitifs la Martinique a vu le nombre de ses exploitations agricoles passer de 8 000 à 3 300. Cette diminution a été particulièrement marquée pour les petites structures. Aujourd'hui, 66 % des 2 994 exploitations agricoles présentent une surface agricole utile, ou SAU, de moins de 5 hectares. L'agriculture couvre désormais 21 % du territoire, soit une diminution de 23 % de la SAU en dix ans. En outre, entre 2013 et 2014, nous avons assisté à une régression de 14 % des cultures légumières, de 6 % des cultures fruitières semi-permanentes et de 30 % des cultures fruitières permanentes

de l'enseignement agricole et une intensification de la politique d'encouragement à l'installation. Mais comment y parvenir quand l'on promet aux potentiels jeunes agriculteurs travaux pénibles et horaires à rallonge, faibles revenus durant leur vie active et retraite aux antipodes de tous les efforts fournis pendant tant d'années ? Selon le rapport de 2016 du Conseil d'orientation des retraites, les prestations de retraite pour une carrière complète s'élèvent à 1 690 euros pour les salariés agricoles et à 710 euros pour les non-salariés agricoles, soit un niveau inférieur à la fois au seuil de pauvreté et à l'allocation de solidarité aux personnes âgées, sachant qu'un non-salarié agricole monopensionné sur deux en outre-mer perçoit une retraite mensuelle inférieure à 333 euros ! Nos

En attendant, peut-être, de meilleures propositions du Gouvernement dans le cadre du prochain projet de loi agricole, sur lequel nous serons extrêmement vigilants, j'ose espérer que cette proposition de loi ira au terme de son cheminement législatif pour une réelle application, rendue plus que nécessaire ! La parole

les agriculteurs sont des passionnés. Ils aiment leur travail. Ils travaillent pour faire progresser leur ferme, leur productivité et la richesse de notre pays. Les agriculteurs, notamment les éleveurs, ont eu des journées, des mois, des années pleines de difficultés : responsabilité sanitaire, responsabilité de vendre leurs produits en essayant de dégager un excédent pour faire vivre leur famille et payer les emprunts. En 2016, ils ont même vendu au-dessous du prix de revient. Je connais bien ces agriculteurs à la retraite, qui ont travaillé sept jours sur sept toute leur vie sur des petites propriétés, qu'ils ont

Si le Gouvernement ne veut pas de ce texte, il a toutefois la responsabilité de respecter le débat démocratique et son expression. Cette proposition de loi, votée à l'unanimité par les députés,

En outre, le texte est parfaitement cohérent avec les engagements de campagne du candidat Emmanuel Macron en faveur de la revalorisation des retraites agricoles. Sur le fond, c'est insultant pour une profession en détresse depuis des années. Pour eux, la situation est intenable. Si je peux Si je peux entendre que le Gouvernement souhaite par cohérence retarder la revalorisation des retraites agricoles pour la faire coïncider avec la réforme globale annoncée des retraites, il n'en demeure pas moins que la situation des agriculteurs de nos territoires en matière de retraite est dramatique. Et c'est encore plus vrai pour les agricultrices, qui, pour une grande part, n'ont pas de statut professionnel ou relèvent du statut de conjointe collaboratrice, lequel ne les couvre pas en l'espèce. Aujourd'hui, nous nous retrouvons autour de la proposition de loi « revalorisation acte II

Voilà Quelle déception, madame la ministre ! Quelle déception de constater que le Gouvernement veut une nouvelle fois jouer de tous les artifices de la procédure parlementaire pour entraver l'adoption définitive de ce texte En déposant deux nouveaux amendements, en apparence favorables aux agriculteurs, vous tentez d'atténuer votre stratégie d'obstruction à ce texte présenté par nos collègues communistes. Mais nous ne sommes pas dupes ! Votre unique objectif est d'empêcher à tout prix un vote conforme du texte adopté à l'unanimité à l'Assemblée nationale. La procédure du vote bloqué soumet la Haute Assemblée à votre souhait d'enterrer au plus vite ce texte. Est-ce cela la démocratie responsable et efficace que vous prônez ? Une démocratie dans laquelle le Parlement serait hors-jeu ? Vous pourriez tout à fait déposer ces amendements dans le cadre d'autres véhicules législatifs et permettre ainsi l'adoption de la revalorisation des petites retraites agricoles à 85 % du SMIC dès cette année. C'est le principal sujet de la proposition de loi ; c'est celui qui nous rassemble ce soir, au-delà des clivages politiques. Il y a une urgence sociale, vous le savez. Repousser l'entrée en vigueur de ce texte reviendrait à nier la précarité de ces hommes et de ces femmes de la terre. Plutôt que de laisser les sénateurs voter la loi en l'état, vous fomentez une nouvelle diversion et vous exercez un marchandage tactique sur le dos des agriculteurs. Ce n'est pas acceptable ! Très en toute logique, nous sommes opposés à ces amendements-postiches, qui, aussi pertinents soient-ils, sont des leurres destinés à fracturer la quasi-unanimité de la Chambre haute, démontrée le 7 mars dernier. Les deux sujets que vous mettez au dernier moment sur la table sont loin d'être sans intérêt pour les agriculteurs. Vous pouvez compter sur nous pour vous rappeler ces bonnes intentions le temps venu. Dans le cas présent, il fallait adopter rapidement ce texte. Vous nous l'empêchez par la procédure du vote bloqué et décevez du même coup l'ensemble du monde agricole et rural, qui nous regarde et soutenait unanimement l'adoption de ce texte sans modification.

vous avez maintenu le recours au vote bloqué, comme vous l'aviez d'ailleurs annoncé à l'issue de nos débats le 7 mars dernier. Vous n'avez pas bougé d'un iota. Vous non plus ! Nous constatons donc une fermeture totale de votre part sur un sujet qui fait pourtant l'objet d'une quasi-unanimité.

également d'ailleurs dans vos projets de loi organique et ordinaire, lesquels visent ni plus ni moins à réduire la place du Parlement dans l'architecture institutionnelle de notre pays Je veux maintenant profiter de l'examen de l'article 1 du présent texte pour évoquer la situation catastrophique des retraités agricoles outre-mer. Les principales raisons de cette situation sont connues des superficies agricoles nettement plus faibles, mais aussi la mise en place tardive du régime de retraite de base, ou encore, pour la retraite complémentaire obligatoire, une assiette de cotisations basée non pas sur le revenu professionnel, mais sur la surface des exploitations pondérée par l'activité. Les outre-mer sont donc doublement défavorisées. Ainsi, à La Réunion, où vivent plus de la moitié des 30 000 agriculteurs retraités d'outre-mer, le montant moyen de la pension était- écoutez bien ! -de 375 euros par mois en 2016. Scandaleux ! Les trois quarts d'entre eux perçoivent un revenu inférieur au seuil de pauvreté, et 25 % perçoivent moins de 100 euros mensuels. C'est la raison pour laquelle il est indispensable, dans un premier temps, de supprimer la condition d'une durée minimale d'assurance en tant que chef d'exploitation. À défaut, toute mesure de revalorisation- aujourd'hui 75 %, demain 85 % du SMIC -risque de rester virtuelle. Bien évidemment, d'autres mesures seraient nécessaires pour revaloriser

Traditionnellement le monde agricole a longtemps été considéré, à tort, comme un milieu d'hommes, en oubliant le rôle central des femmes, assumant souvent dans l'ombre une bonne partie des tâches de la ferme. De nos jours, alors que le métier d'agriculteur et d'agricultrice a beaucoup évolué et impose des contraintes très lourdes, les inégalités, notamment lors du départ à la retraite, subsistent, en particulier pour les femmes. Si les femmes ont depuis toujours joué un rôle crucial dans la vie des exploitations agricoles, celui-ci n'a pas toujours été reconnu comme tel. Du fait de leur statut de conjointe ou d'aide occasionnelle, elles restent minoritaires en tant qu'agricultrices à part entière. Les agricultrices qui réussissent à avoir des terres obtiennent bien souvent les plus petits lots lors des ventes. Il est

pour reconnaître une évolution urgente du montant des pensions de retraite : nous ne

Aujourd'hui, nous sommes de nouveau placés devant ce choix. Et, de nouveau, alors que les sénateurs sont quasiment unanimes, vous ne voulez pas de l'adoption de ce texte.

Comme cela a été dit au cours du débat sur le recul du trait de côte, allons-nous enfin sortir de nos circonvolutions habituelles qui, sous des prétextes toujours renouvelés, nous empêchent de régler des situations humaines urgentes ? Allons-nous cesser de remettre à plus tard, sous prétexte d'un mieux, ce que nous pouvons faire de bien ici et maintenant ?

étant, n'ayant pas une pensée suffisamment complexe, je vous propose de nous en tenir à la réalité des faits, lesquels ont une fâcheuse tendance à être têtus

La réalité, c'est celle aussi d'associations, de syndicats, qui se mobilisent pour dire qu'il n'est pas possible que les retraités agricoles vivent sous le seuil de pauvreté : ils se sont sentis trahis par l'attitude du Gouvernement le 7 mars dernier.

La réalité, c'est que votre gouvernement a choisi de privilégier les 330 000 contribuables assujettis à l'ISF, au détriment des retraités agricoles, pour un rapport

aussitôt suivis par les mots « pénibilité », « préjugés » et « invisibilité », surtout quand il s'agit des femmes agricultrices. Nous avons abordé à cette occasion, outre le statut économique critique des agricultrices, la question de la parité dans les instances dirigeantes du monde agricole, la question du statut juridique de la femme conjointe ou collaboratrice d'agriculteur. Marlène Schiappa, qui représentait le Gouvernement lors de ce débat, s'est dite consciente de la situation et particulièrement concernée. Quoi de plus normal, me direz-vous, pour la secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes ? Mais permettez-moi, mes chers collègues, de dénoncer le scénario ubuesque que nous vivons une fois de plus aujourd'hui. Au-delà de tous les aspects antidémocratiques qui ont été déjà dénoncés sur le recours au vote bloqué, voilà un gouvernement qui, selon les dires de Marlène Schiappa, attentif et sensible à une situation, mais refuse de prendre en compte notre proposition, laquelle permettrait justement de revaloriser la pension des femmes agricultrices particulièrement malmenées. J'avoue que ce double langage est insupportable ... Notre proposition de loi a justement pour but de répondre à la question des faibles revenus, aux retraites insignifiantes, à la reconnaissance du travail de ces femmes. La refuser aujourd'hui, c'est concrètement refuser de prendre en compte la situation des femmes agricultrices. Une fois de plus, dans une situation où le président Macron a affirmé vouloir faire de l'égalité entre les femmes et les hommes une grande cause nationale, les mesures concrètes ne suivent pas. On pourrait s'amuser à plagier une célèbre chanson et fredonner « Paroles, paroles, paroles », si le contexte n'était pas aussi dramatique ! Madame la ministre, j'aimerais vraiment savoir comment le Gouvernement entend répondre précisément aux problématiques des femmes agricultrices sans permettre la revalorisation des pensions agricoles

est une nécessité pour répondre à une urgence sociale. Non, les retraites des agriculteurs ne sont pas comparables avec les autres retraites ni dans leur niveau ni dans leurs modalités de calcul. aucun argument technique pour attendre qu'elles soient abordées dans le cadre de la réforme générale des retraites prévue en 2020. La retraite moyenne d'un non-salarié agricole, tous bénéficiaires confondus, s'élève aujourd'hui à 766 euros par mois, contre 1 800 euros pour l'ensemble des Français, soit un niveau inférieur

Dans les modalités de calcul des pensions, il existe, là aussi, des différences importantes avec le régime général : pour le monde agricole, l'ensemble de la carrière est pris en compte, alors que, pour les salariés, seules les vingt-cinq meilleures années la Drôme, en 2016, le montant moyen de la pension de retraite d'un non-salarié agricole pour une carrière complète était de 758 euros par mois. Mais les carrières sont, vous le savez, souvent courtes et hétérogènes : moins de 30 % des anciens exploitants justifient d'une carrière complète et moins de la moitié bénéficient

dès 2018, comme nous le proposons aujourd'hui. Hommes ou femmes, cultivateurs ou éleveurs, tous les agriculteurs retraités témoignent des mêmes difficultés : une vie de dur labeur pour une retraite de misère ! Cette situation est vécue comme une injustice. Madame la ministre, il y a urgence à à soutenir le monde agricole. Ce monde contribue à nourrir la France, à développer nos terroirs, à entretenir nos paysages et à maintenir la vie dans nos territoires. Oui, l'urgence sociale et la précarité vécue par des milliers d'anciens paysans ne sont pas acceptables et ne peuvent attendre 2020. L'amélioration des recettes fiscales doit permettre au Gouvernement de trouver, au titre de la solidarité nationale, les 350 millions d'euros nécessaires qui pourraient changer le quotidien de milliers de retraités agricoles et corriger un peu les injustices qui caractérisent ce régime de retraite.

de retraite équivalente à 85 % du SMIC. Aujourd'hui, comme il y a quelques semaines, le Gouvernement se refuse à cette revalorisation. La revalorisation de ces pensions a trait à de multiples enjeux. Des enjeux sociaux tout d'abord, puisque la pension d'un retraité agricole est de 766 euros en moyenne, soit en dessous du seuil de pauvreté. Un retraité agricole sur trois a même une pension de retraite inférieure à 350 euros. Mais cette revalorisation est aussi un enjeu de genre puisque, aujourd'hui, les femmes bénéficiant de ce régime touchent des retraites deux fois et demie moins élevées que celles de leurs collègues masculins, soit environ 500 euros à 550 euros mensuels. Enfin, il s'agit d'un enjeu territorial qu'en outre-mer les retraites descendent parfois jusqu'à 100 euros par mois ! Vous en conviendrez, ces rémunérations sont iniques et indignes, en particulier pour des travailleurs qui ont connu un labeur harassant tout au long de leur vie professionnelle. Par ce refus doctrinal de revaloriser les pensions des plus modestes, le Gouvernement fait preuve d'un mépris sans nom envers nos concitoyens les plus démunis du monde rural. Pire encore, il accroît la fracture sociale et territoriale entre villes et campagnes. Gouverner, pourtant, ce n'est pas diviser. Ce n'est pas non plus maintenir dans la précarité. Nous avons certes compris que ce gouvernement avait plus à coeur les intérêts des patrons du CAC 40. Nous espérons cependant un geste pour ces retraités agricoles qui le méritent tout autant, si ce n'est

chers collègues, nous sommes de nouveau devant un abus de droit du Gouvernement qui cherche par tous les artifices réglementaires à nous imposer le vote bloqué. La démocratie est en danger Ce passage en force est d'autant plus regrettable qu'il constitue la seule réponse du Gouvernement à l'égard d'une profession en grande difficulté dans l'Hexagone, mais aussi dans les outre-mer. Reporter ainsi l'application des dispositions de cette proposition de loi à 2020 est, à l'évidence, une forme de mépris vis-à-vis des travailleurs de la terre qui, après toute une vie de dur labeur, ont des retraites inférieures au seuil de pauvreté. Ils vivent dans la misère, madame la ministre ! Ce gouvernement est manifestement sourd.

Au mois de mars dernier, le journal a consacré un article à la situation des agriculteurs, particulièrement au taux de suicide dans la profession. La situation est triste. Vous comprendrez que les mesures de justice et d'équité concernent également les outre-mer,

d'une profession qui, à force de sacrifices, participe à notre alimentation en privilégiant les circuits courts et en préservant nos réserves foncières. Il est important que l'on puisse sauver des agriculteurs puisse sauver des agriculteurs du suicide, de la misère. Il faudrait que vous soyez vigilants et à l'écoute de ces personnes qui souffrent. Certains d'entre eux ont fait le déplacement pour entendre, pour voir, pour écouter, pour comprendre d'où vient le mal ! Aussi, en toute conscience, je porte mon soutien indéfectible à l'ensemble des agriculteurs. Madame